Mes chers collègues, en raison de la réunion de la conférence des présidents de ce jour, et en accord avec le Gouvernement, nous pourrions suspendre nos travaux à l'issue de la séance de questions d'actualité au Gouvernement et les reprendre à dix-huit avec la poursuite de l'examen du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. Il n'y a pas d'observation ? ... Il en est ainsi décidé. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour un État au service d'une société de confiance

Monsieur le président, monsieur le président de la commission spéciale, madame le rapporteur, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis dix mois maintenant, la France est engagée dans un mouvement de transformation profond : transformation économique, transformation fiscale, transformation écologique. Dans notre pays, le service public occupe une place centrale et suscite beaucoup d'attentes chez nos concitoyens. L'administration doit donc être dans ce moment un moteur de transformation, un moteur de progrès. Pourtant, nous le savons tous, notre pays est frappé d'un paradoxe : les Français aiment leurs services publics, mais ils critiquent et parfois rejettent leur administration. Un chiffre suffit à illustrer cette réalité : la satisfaction des usagers du service public est supérieure de 30 points à l'image qu'en ont les Français dans leur ensemble. Parfois aussi ce sont les agents publics qui doutent de leur propre administration et des moyens qui sont mis à leur disposition. Le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance entend donc libérer les énergies et les initiatives au sein de notre administration. Il porte une vision positive et bienveillante du service public et des agents qui le font vivre. Il leur donne les moyens de jouer un rôle nouveau dans la vie des Françaises et des Français. C'est pourquoi nous avons voulu affirmer deux grands principes dans ce texte : d'abord, une administration qui conseille avant de sanctionner ; ensuite, une administration qui simplifie plutôt que de complexifier. Ces principes sont indispensables, car ce sont eux qui montrent le cap et les priorités du texte que nous vous présentons. Mais ce projet de loi apporte surtout des réponses très concrètes aux usagers et aux agents publics, en combinant mesures générales et mesures expérimentales. Je m'arrêterai d'abord sur le premier pilier de ce texte, celui de la confiance. C'est le principe même du droit à l'erreur que ce projet de texte consacre, pour les entreprises comme pour les particuliers. Vous le savez, le droit à l'erreur était un engagement du Président de la République. Demain, cette révolution sera à l'oeuvre : dans le cadre d'une déclaration à l'administration ou d'un contrôle, l'usager de bonne foi pourra revendiquer un « droit à l'erreur » et l'administration le dispensera de pénalité. Ce principe ne souffrira que d'exceptions de bon sens. Pour l'administration fiscale et douanière, le texte comporte une disposition supplémentaire puisque, s'agissant des intérêts de retard, le principe qui vaudra sera celui de la « faute avouée à moitié pardonnée », avec des intérêts divisés par deux lorsque la rectification viendra du contribuable lui-même. Le projet de loi consacre également pour nos entreprises des mesures qui découlent directement de cette philosophie et qui faciliteront leurs relations avec l'administration. J'insisterai sur trois d'entre elles. il crée un « droit au contrôle », pour que chaque entreprise puisse s'assurer qu'elle est bien en règle et bénéficier des conclusions de ce contrôle comme d'un rescrit. Deuxièmement, il instaure une limitation de la durée de contrôle pour les PME, sous forme expérimentale, pour que cette durée ne puisse dépasser neuf mois sur trois ans, soit un quart du temps de l'entreprise. prévoit la création d'un avertissement avant la sanction par l'inspection du travail, parce qu'avant de donner un carton rouge, l'administration doit pouvoir adresser un carton jaune à l'entrepreneur de bonne foi. Le Gouvernement a donc tenu à intégrer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le travail et les PME, mais aussi des dispositions sectorielles, pour fluidifier davantage le fonctionnement de certaines activités. Nous avons ainsi travaillé avec le ministre de l'agriculture pour intégrer des dispositions spécifiques relevant de son champ de compétence. Nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir dans nos débats. Ce projet de texte prévoit également des mesures pour les particuliers, qui pourront bénéficier du droit à l'erreur et du droit au contrôle en plus d'autres mesures spécifiques ; je pense, notamment, au droit à la rectification lors de la réclamation d'indus dans le champ social. Enfin, ce texte vise aussi à offrir aux agents de la fonction publique la possibilité d'établir le dialogue avec les usagers. Bien souvent, ils le voudraient, mais ils ne disposent pas des outils pour cela.

Le second pilier de ce texte sur lequel je souhaite m'arrêter un instant est celui de la simplicité. Il s'agit, pour les usagers du service public, d'une nécessité absolue. Pour la comprendre, on peut évoquer un chiffre éloquent : la France occupe le cent quinzième rang- sur cent quarante -en matière de complexité administrative.

Ensuite, l'adaptation des horaires d'ouverture des services publics aux habitudes de vie des Français, conformément à l'engagement du Président de la République. Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, s'est ainsi proposé d'expérimenter cette adaptation dans deux juridictions de taille importante. Enfin, un autre engagement trouve ses premières traductions dans ce texte : celui du « zéro papier » d'ici à 2022, avec la dématérialisation de l'ensemble des déclarations administratives. Des premières annonces ont été faites à l'occasion du comité interministériel de la transformation publique qui s'est Ce texte de loi consacre, par exemple, l'extension par expérimentation du principe « dites-le-nous une fois », qui devient en réalité le principe « dites-le-nous une fois, mais une fois pour toutes » Pour promouvoir la confiance et la simplicité dans les relations entre les citoyens et l'administration, nous devons par ailleurs revoir notre rapport à la norme et à la loi, la manière dont nous la concevons et dont nous la faisons connaître. Ce texte se fixe donc pour ambition de changer les habitudes de l'administration, qui se contente trop souvent d'opposer à nos concitoyens l'adage : « Nul n'est censé ignorer la loi ». Lorsque la loi devient trop complexe, qui peut vraiment la connaître ? Le projet de loi comporte ainsi de nombreuses mesures qui permettront de repenser en profondeur la fabrique et l'application des lois et des règlements. Le texte s'efforce ainsi d'adapter la norme à la diversité des territoires, que vous connaissez tous, mesdames, messieurs Cette adaptation est rendue possible, en particulier par l'expérimentation, qui permet de tester la pertinence d'une nouvelle norme, son efficacité, avant de la généraliser ou bien d'y renoncer. Ce projet de loi met en oeuvre bien d'autres outils sur lesquels je souhaite appeler votre attention. D'abord, la transparence sur les centaines de circulaires qui produisent des effets sur nos concitoyens et sont inconnues d'eux. Ensuite, la lutte contre la surtransposition des directives européennes. Je pense, par exemple, à la suppression du rapport de gestion pour toutes les petites entreprises, ce qui représente une journée de travail en moins pour 1,3 million de petites entreprises, soit une économie de 270 millions d'euros. Enfin, l'inversion complète de notre manière de faire la loi dans certains secteurs nous souhaitons, par exemple, expérimenter dans le domaine de la construction une nouvelle obligation qui soit une obligation de résultat et non plus une obligation de moyens. Je veux dire maintenant quelques mots de la méthode singulière qui a conduit à l'élaboration de ce texte. Il s'agit d'abord d'une loi qui a été coconstruite avec les différents membres du Gouvernement, avec des experts comme le conseiller d'État Thierry Tuot et, bien évidemment, avec le Parlement. La première lecture à l'Assemblée nationale s'est tenue dans un état d'esprit d'ouverture et nous souhaitons nous inscrire dans la même logique au Sénat. Vos travaux en commission ont déjà permis d'améliorer substantiellement le projet de texte, sur la forme, avec de nombreuses améliorations légistiques et rédactionnelles, mais également sur le fond. Je pense, par exemple, à la précision apportée à l'article 2 sur le droit à l'erreur cet article prévoit désormais que l'administration est tenue d'inviter un usager à régulariser sa situation dès qu'elle s'aperçoit de l'erreur, ce qui permettra de rendre ce droit plus effectif. On peut également citer le dispositif de l'article 4, pour lequel vous avez précisé les conditions dans lesquelles pouvait être accordée la réduction des intérêts de retard en matière douanière. pour la première fois, la procédure dite de « législation en commission » a été utilisée sur certains articles de ce texte, ce qui nous permettra de nous concentrer en séance sur les articles les plus importants. Dans cette nouvelle phase de débats, nous serons le plus à l'écoute possible de vos propositions. C'est aussi une loi qui s'inspire des bonnes pratiques étrangères. Je vous en donne quelques exemples. Les Pays-Bas pratiquent depuis longtemps ce que nous appelons la relation de confiance entre les entreprises et l'administration fiscale le principe de la suppression de deux anciennes normes pour une nouvelle norme créée est appliqué en Grande-Bretagne ; de la même manière, en ce qui concerne la lutte contre la surtransposition, notre projet s'inspire des mesures mises en oeuvre en l'Allemagne et dans d'autres pays. pays. Pour conclure, ce projet de loi devra faire l'objet d'un suivi renforcé. Le Gouvernement s'efforcera de suivre précisément l'application de la loi à travers la publication des décrets, bien les résultats des différentes expérimentations que ce projet contient et en suivant la mise en application concrète des mesures qui auront été adoptées. Nous serions heureux que les parlementaires, notamment ceux de la Haute Assemblée, prennent part directement à ce suivi opérationnel. même avec un texte que je crois être de qualité et qui sera enrichi de vos propositions, nous ne devons pas nous arrêter là. En effet, sans vouloir me montrer décourageant, même si le Parlement adopte ce texte, même si nous le mettons rapidement en oeuvre, nous n'aurons fait qu'une toute petite partie du chemin. Les changements les plus importants ne sont pas dans les textes, ils sont dans les têtes. À cet égard, pour ce qui concerne la fonction publique, la formation de nos agents est capitale. Le Gouvernement sera au rendez-vous : dans le cadre du Grand plan d'investissement, 1,5 milliard d'euros ont ainsi été identifiés et dédiés au financement de la formation des agents publics pour accompagner la transformation des services publics. Voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce qui constitue pour nous la première pierre du programme Action publique 2022. Cet acte I de la transformation publique témoigne de l'ambition qui est celle du Gouvernement de remettre la confiance au coeur des relations entre l'administration et les usagers. Je souhaite que les débats qui s'ouvrent puissent nous permettre d'aller encore plus avant sur ces différents sujets. La parole est

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, je pourrais me contenter de vous dire que ce texte, après avoir suscité beaucoup d'attentes, a beaucoup déçu, mais cela ne serait pas faire honneur au travail accompli par notre commission. Nous avons en effet choisi de nous départir de tout et d'aborder ce projet de loi de manière constructive, avec la volonté de le rendre plus opérant et, surtout, de lui donner une cohérence qui lui faisait défaut. L'article 2 crée deux dispositifs : tout d'abord, un « droit à l'erreur », au bénéfice de tout usager qui méconnaîtrait involontairement, et pour la première fois, une règle applicable à sa situation ensuite, un « droit au contrôle », auquel l'administration est tenue de répondre dans un délai raisonnable, et dont les conclusions sont opposables. Ces deux nouveaux dispositifs sont supplétifs par rapport aux « droits à l'erreur » spécifiques. Si l'ensemble manque de précision et est dépourvu d'étude d'impact, il n'y a pas de raison de principe de s'y opposer. La commission spéciale a toutefois adopté une série d'ajustements pour préciser le dispositif, l'ouvrir davantage et le rendre plus incitatif. Je signale, en particulier, l'extension du bénéfice du droit à l'erreur aux collectivités territoriales dans les relations qu'elles entretiennent avec l'État. Au-delà de l'article 2, plusieurs dispositions entendent rétablir un lien de confiance entre l'État et la société. Ainsi en est-il de l'article visant à interdire aux administrations de l'État de recourir à un numéro surtaxé dans leurs relations avec le public. Cela évitera le sentiment d'amertume que peuvent ressentir certains de nos concitoyens lorsqu'ils attendent d'être mis en relation avec un interlocuteur alors que chaque minute est facturée. Par ailleurs, la commission spéciale a adopté un amendement modifiant la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, en vue d'exclure les responsables locaux du champ d'application de ses dispositions relatives aux relations entre les représentants d'intérêts et les responsables publics. L'extension de ces dispositions aux élus locaux n'aurait, à mon sens, qu'une faible valeur ajoutée. En effet, l'objectif premier du répertoire numérique est de faire la transparence sur l'influence des représentants d'intérêts relativement à l'élaboration de la loi et du règlement national-les national-les relations quotidiennes qui se nouent sur les territoires n'en font assurément pas partie. Cet avis est partagé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui m'a alertée sur le sujet, confirmant des inquiétudes déjà exprimées sur son incapacité à faire face à ce surcroît d'activité au 1 juillet 2018. S'agissant des dispositions fiscales du texte, et au risque de tempérer l'enthousiasme affiché par le Gouvernement, je rappelle que le droit à l'erreur existe depuis bien longtemps dans ce domaine : le contribuable est toujours présumé de bonne foi et les majorations ne peuvent être appliquées que si l'administration apporte la preuve d'une intention frauduleuse. Les articles qui prévoient la diminution de l'intérêt de retard en cas de régularisation n'ont donc rien à voir avec un « droit à l'erreur ce sont des mesures incitatives au civisme fiscal. J'insiste sur ce point : l'intérêt de retard n'est pas une sanction, c'est le « prix du temps ». C'est pour cela que la commission n'a pas souhaité qu'il soit entièrement supprimé. supprimé. Le texte contient tout de même quelques dispositions substantielles en matière fiscale. La première, la « garantie fiscale », provient non pas du Gouvernement mais de nos collègues députés. Elle vise à inscrire dans la loi que tout point examiné lors d'un contrôle fiscal et n'ayant pas fait l'objet d'un redressement serait considéré comme tacitement validé par l'administration. Cela semble être la moindre des choses, mais il se trouve que ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'autre disposition fiscale substantielle est la relance de la « relation de confiance ». Lancée en 2013, cette expérimentation consiste à valider en amont les options fiscales d'une entreprise plutôt qu'à les sanctionner en aval par un contrôle fiscal. La commission a précisé l'habilitation prévue à l'article 7, qui était trop vague, afin de préserver l'esprit initial de la relation de confiance, c'est-à-dire en donnant la priorité à un accompagnement continu des entreprises dans leurs obligations déclaratives. Cela dit, fondamentalement, quand on parle d'amélioration des relations avec l'administration fiscale ou encore de passage d'une logique de contrôle et de sanction à une logique de conseil et d'accompagnement, il s'agit avant tout d'une question de changement culturel et d'organisation bien plus que d'une question législative. Monsieur le secrétaire d'État, c'est à votre gouvernement d'agir ! Inutile de vous dire que le chemin sera long ... J'en viens aux dispositions touchant aux affaires sociales. Elles visent notamment à développer la médiation au sein des URSSAF, du régime agricole et des branches Vieillesse et Famille du régime général. Dans le cadre de la procédure de législation en commission, la commission spéciale a adopté plusieurs amendements visant à préciser ces dispositions, et à éviter que celles-ci n'entravent l'équilibre et le bon fonctionnement des dispositifs déjà existants. L'Assemblée nationale avait introduit un article créant une forme de « super-médiateur », habilité à résoudre les différends entre les entreprises et les administrations. La commission a supprimé cette disposition à titre conservatoire, car elle semble inaboutie, voire source de confusion. Le texte prévoit aussi d'expérimenter un cadre dérogatoire au droit du travail pour permettre la mise en place de prestations de relayage des proches aidants. La commission a choisi de laisser sa chance à cette disposition, après quelques modifications pour la rendre plus réaliste. Elle a aussi adopté un article visant à moduler le montant de l'annulation des exonérations de cotisations sociales

tout en adhérant aux grands principes du texte, la commission spéciale a cherché à le recentrer sur son objet initial- c'est-à-dire sur l'amélioration des relations entre le public et l'administration

C'est ainsi qu'en matière de rescrit, dont elle partage la philosophie, la commission est revenue sur sa généralisation à toute l'administration, à défaut de précisions suffisantes sur la portée de la réforme envisagée, et qu'elle a également simplifié l'expérimentation d'un dispositif voisin en matière juridictionnelle pour sécuriser les grands projets sans surcharger les tribunaux administratifs. En matière d'information et de sécurité juridique des usagers, nous avons, d'une part, élargi à certaines notes l'obligation de publicité des instructions et circulaires qui conditionne leur prise d'effet et, d'autre part, renforcé le droit au certificat d'information : ce droit sera désormais ouvert à tout usager exerçant ou souhaitant exercer une activité, avec obligation pour l'administration de l'orienter, si besoin, vers d'autres interlocuteurs administratifs dans le mois suivant sa demande et, surtout, de lui répondre, sur le fond, dans les trois mois. En outre, si la création de référents uniques est une bonne idée, l'application de la mesure aux maisons de services au public nous a semblé inopportune tant ces structures sont diverses : il vaut mieux s'en remettre, en la matière, au terrain. La commission a en revanche approuvé l'expérimentation d'une limitation de la durée cumulée des contrôles administratifs sur les PME.

En matière agricole, la commission s'est assurée que les transferts de compétences des chambres départementales d'agriculture vers les chambres régionales ne seraient expérimentés qu'avec l'accord des intéressés. Elle a par ailleurs maintenu la suppression des mesures d'allégement sur le contrôle des structures agricoles, mesures qui faisaient l'unanimité contre elles. Dans le secteur de la construction, la commission a accueilli favorablement la possibilité de déroger, par voie d'ordonnances, à certaines règles de la construction, mais sous réserve de limiter le délai d'habilitation à douze mois, à douze mois, et après avoir reçu du Gouvernement l'assurance qu'il n'était pas question de revoir à la baisse le niveau des exigences et des contrôles. Je pense, notamment, à tout ce qui concerne la sécurité. En matière d'enseignement supérieur, nous avons approuvé la possibilité d'expérimenter, là aussi par ordonnance, de nouvelles formes de regroupement d'établissements, mais en limitant cette fois l'habilitation à six mois, pour une mise en oeuvre rapide. Concernant la participation du public aux projets qui ont une incidence sur l'environnement, la commission s'est opposée à l'idée de remplacer, même à titre expérimental, l'enquête publique par une simple procédure de consultation par voie électronique pour certains projets agricoles, au motif, en particulier, que cette enquête publique en favorise l'acceptabilité et que s'en passer pourrait se révéler contre-productif pour les agriculteurs eux-mêmes. Pour sécuriser et accélérer les projets, nous avons en revanche prévu de réduire de quatre à deux mois le délai de recours des tiers contre les décisions administratives relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement. maintenant, la commission adhère à la philosophie des mesures de simplification proposées en matière d'énergies marines renouvelables ou de géothermie, mais a également souhaité réduire la durée, voire le champ des habilitations demandées par le Gouvernement. Nous avons aussi clarifié et mieux encadré le droit reconnu à tout producteur ou consommateur de faire réaliser son raccordement au réseau électrique par des entreprises agréées. Enfin, la commission a jugé nécessaire de réduire le nombre de rapports sur un texte qui n'en comptait pas moins d'une cinquantaine. À l'exception de l'évaluation des diverses expérimentations, indispensable avant d'envisager une généralisation éventuelle, ces rapports, à supposer qu'ils soient effectivement remis, ne permettent en effet que très rarement de résoudre les problèmes identifiés. En l'espèce, les demandes de rapports que nous avons supprimées procédaient surtout de la volonté d'étayer « un dispositif d'évaluation renouvelé » de la loi, mais sans contenu réel ... Vous l'aurez constaté, mes chers collègues, malgré nos efforts, il s'agit encore d'une loi relativement « fourre-tout », dont l'intention est souvent louable, mais dont la portée est parfois limitée, voire déclamatoire. J'ajoute que certaines des procédures qu'elle crée, ou qu'elle généralise, appelleront sans doute des moyens humains et matériels ou des actions de formation supplémentaires, dimension que le texte n'aborde pas. Nous allons débattre sur tous ces sujets et voir si l'avis de la commission sera suivi ou amendé. Cette loi ne révolutionnera pas la relation entre l'usager et son administration, mais elle va tout de même dans le bon sens. Puisse désormais cette culture nouvelle de la confiance passer du slogan à la réalité ... Mes chers

Ce projet de loi, j'ai envie d'y croire. Comme j'ai eu l'occasion de le dire en commission, j'en partage en grande partie la philosophie. Vous prolongez en quelque sorte le travail initié par MM. Warsmann et Mandon en leur temps. Chaque élu rêve d'une société où nos concitoyens n'auraient aucun problème à dialoguer avec leur administration. Nous en sommes loin aujourd'hui ! Votre texte propose donc l'approbation d'une stratégie nationale d'orientation de l'action publique. Cette stratégie vise à poser les conditions d'une confiance retrouvée du public dans l'administration. Le titre Idu projet de loi consacre en effet un droit à l'erreur, notamment en matière fiscale, avec une réduction des intérêts de retard en cas de dépôt spontané par le contribuable d'une déclaration rectificative. Sera aussi expérimenté, au sein de l'administration, un référent unique, pour chaque usager, afin de faciliter les démarches dans le cadre de procédures ou dispositifs particuliers. Le titre II ambitionne une action publique modernisée, simple et efficace en introduisant, à titre expérimental, la faculté pour les entreprises de ne pas communiquer à une administration des informations déjà détenues par celle-ci dans le cadre d'un traitement automatisé. Le texte prévoit enfin le « relayage » au domicile, qui permet d'assurer la continuité de l'accompagnement d'une personne âgée en perte d'autonomie, chez elle, pendant plusieurs jours successifs. de loi, monsieur le secrétaire d'État, vise à simplifier, mais il se révèle pourtant complexe et divers- « fourre-tout », disent certains. C'est souvent l'une des conséquences des bonnes intentions en la matière ; je serais bien ingrat de trop vous le faire remarquer puisque le groupe socialiste et républicain portera lui-même des amendements de nature assez diverse. J'ai néanmoins déposé, au nom de mon groupe, un amendement de modification du titre du projet de loi qui, au vu de ce qui précède, me paraît un peu pompeux. Pour vous ôter tout doute quant à ma bonne foi, je vous ferai un compliment, monsieur Dussopt : votre projet de loi, comporte, c'est suffisamment rare pour être souligné dans le quinquennat Macron, assez peu de chiffons rouges pour l'homme de gauche que je suis.

Mais la confiance, pour exister, doit être partagée par tous les maillons de la chaîne. Il me semble, monsieur Dussopt, que c'est là que le bât blesse. Les fonctionnaires ne font aujourd'hui pas totalement confiance à leur gouvernement. Vous leur demandez, avec ce projet de loi, de fournir un travail toujours plus important. Dans le même temps, ils dénoncent une baisse des moyens qui leur sont consacrés. Votre volonté de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires en constitue une illustration édifiante.

ne dispose pas des moyens qui devraient lui être consacrés. Au fond, monsieur le secrétaire d'État, le conseil n'exclut pas le contrôle. Et votre administration, avec moins de moyens, devra faire les deux. La simplification pour les uns se traduira nécessairement par du travail pour les autres. L'autre reproche que je souhaiterais formuler sur ce projet de loi est le caractère parfois trop général des dispositions législatives qui nous sont proposées. C'est sur la base de principes souvent très généraux qu'une très large délégation est accordée au Gouvernement : douze ordonnances, quinze expérimentations ! Un parlementaire qui veut contribuer concrètement à l'action publique peut rester sur sa faim, notamment dans le contexte de révision constitutionnelle que l'on connaît. D'autres points divers du texte méritent réflexion. Je pense, notamment, à la fin des numéros surtaxés pour joindre les services de l'État, qui représentaient une aberration pour nos concitoyens recherchant une aide précise et directe. Cette fin nécessaire des numéros de téléphone surtaxés constitue un bon point, car tout ne se passe pas sur internet, même en 2018-

chers collègues, en matière de transparence comme en matière du droit du travail ! Nous abordons donc, monsieur Dussopt, l'examen de ce texte dans un esprit ouvert, mais avec toute la vigilance nécessaire.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission spéciale, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui un texte important pour la refondation des relations entre l'administration et les usagers.

de logiciel et même de culture, à tous les échelons de l'administration. Cela fait des années que nous essayons d'instaurer une culture de la confiance entre les administrations, les citoyens et les entreprises. Cela fait des années que nous essayons de rompre avec la maxime classique de La Rochefoucauld selon laquelle la bonne administration « doit être un mystère caché aux regards du peuple

Je veux le souligner ici, la volonté d'ouverture du Gouvernement a été admirablement accompagnée, voire parfois précédée, par le Sénat. la commission spéciale sénatoriale- c'est l'honneur de son président, Jean-François Husson, et de ses rapporteurs, Pascale Gruny et Jean-Claude Luche -a été à l'initiative de nombreux amendements pragmatiques de clarification, de précision ou, tout simplement, de suppression des dispositions les moins pertinentes. Je regrette seulement que cette volonté d'efficacité et de bon sens ait peut-être été poussée un peu loin sur la partie du texte relative à l'évaluation,

De même, la chasse légitime à l'incompétence négative menée par la commission a conduit à vider de leur substance plusieurs dispositions du texte issu de l'Assemblée nationale, notamment l'article 10, portant sur la généralisation du rescrit, qui contenait des avancées intéressantes. Néanmoins, nous pouvons dire que l'action conjointe du Gouvernement, du Sénat et de l'Assemblée nationale a conduit à un texte plus robuste et plus réaliste, bien qu'il reste en deçà du choc de confiance annoncé.

Je vous présenterai pour ma part deux amendements visant à mieux prendre en considération la situation particulière des PME et des TPE dans leurs rapports avec l'administration. Les grandes entreprises ont davantage de moyens pour traiter la complexité ; nous devons donc redoubler d'attention pour les plus petites, qui n'en ont pas de tels, mais qui sont si essentielles à notre économie. Je pense également à des problèmes plus structurels, ceux de l'inflation et de l'instabilité normatives, une composante essentielle du manque de confiance des usagers envers l'administration.

Alors que les débats sur le projet de révision constitutionnelle commencent, je crois que cette problématique gagnerait à être abordée plus sereinement, dans l'idée d'un meilleur pilotage de l'activité normative, sans remettre en cause les droits constitutionnels du Parlement. La confiance entre le Gouvernement et le Parlement est aussi essentielle à une République moderne que celle qui existe entre l'administration et l'usager. Enfin- troisième point d'incertitude sur lequel vous devrez faire preuve de courage et d'ambition, ce texte appelle de nombreuses expérimentations, de nombreuses habilitations, de nombreux décrets d'application et exigences d'évaluation. En un mot, une grande responsabilité pèse sur le Gouvernement et sur les administrations pour faire de ce projet de loi et de ses grands principes une réussite concrète et tangible. L'adoption de ce texte doit être non pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle logique pour l'administration, qui sera largement responsable de son échec ou de son succès. L'administration devra mériter la confiance que le législateur et l'ensemble des Français placeront en elle pour simplifier et améliorer le quotidien Le droit à l'erreur était une promesse de campagne du Président de la République, une campagne placée sous le signe de la confiance ; mais la confiance ne se décrète pas, elle se construit patiemment, brique par brique, elle se mérite au quotidien. Si, pour paraphraser Gustave Le Bon, ce sont les bâtisseurs de confiance qui mènent l'histoire, le groupe Les Indépendants - République et Territoires participera volontiers à cet effort pour construire une France réconciliée, plus confiante et plus unie.

m'amène à formuler un certain nombre de remarques, je dirais même de réticences, aussi bien sur le fond que sur la forme. Tout d'abord, sur le fond, il y a des dispositions qui relèvent véritablement de la logique du droit à l'erreur, mais,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission spéciale, cher Jean-François Husson, madame, monsieur les rapporteurs, chers Pascale Gruny et Jean-Claude Luche- vous avez fait preuve d'une écoute fort appréciable que je tiens à saluer -, mes chers collègues,

avons qualifié de texte attrape-tout, à l'image de nombreuses lois dites de simplification que le Parlement a eu à examiner sous chaque législature Que dire de ce texte qui peut s'apparenter à un contresens législatif, puisqu'il nous demande, à nous, législateur, de consacrer, sur 65 articles, pas moins de 12 demandes d'habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances Jusqu'à aujourd'hui, la relation de confiance entre les usagers et leur administration a su s'instaurer autour de principes généraux applicables au service public, comme la continuité, l'égalité, l'accessibilité, mais aussi la neutralité et la laïcité. C'est ainsi que s'est construit le service public à la française, sous l'égide du Conseil d'État. Dans le respect de ces principes, le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen accueillait donc favorablement ce projet de réforme, au vu de l'impérieuse nécessité d'une modernisation de l'action publique, aussi bien dans ses finalités que dans ses procédés.

la société évolue, tout comme notre environnement économique et social. La définition même de l'intérêt général, que l'on sait contingente, ne saurait rester figée. Il est donc parfaitement cohérent que l'administration évolue elle aussi, notamment dans ses relations avec le public. Dans ce cadre, nous saluons la décision de la commission spéciale d'étendre ce dispositif à l'ensemble des usagers : citoyens, entreprises et collectivités territoriales. pour plus de proximité entre l'administration et son public, d'un droit à la régularisation, communément présenté comme un droit à l'erreur, qui permet à un usager de commettre une erreur de bonne foi, à condition qu'elle soit rectifiée et que cela soit la première occurrence,

et à garantir une meilleure information correspond à notre demande et à ce que l'on peut attendre d'un texte de confiance entre la société et son administration. Il convient de rappeler ici le rôle central de l'administration comme régulateur de la société, comme acteur du pacte social et de la préservation de l'intérêt général. Il est donc regrettable que ce projet de loi conduise à légiférer sur des sujets si divers,

Après les atermoiements du Gouvernement sur les retraites agricoles, nous demandons que cette question importante ne soit pas traitée au détour d'un article noyé dans la masse, mais fasse l'objet d'une discussion à part entière. Tout aussi diluées dans le flot de ces nombreux articles, des dispositions introduites par le Gouvernement modifient la loi de 1905 et le principe de séparation des Églises et de l'État, et ce de façon non marginale. La loi de 1905 a fait de la France un État laïque, et ce principe fondateur a, dans notre République, L'article 2 de cette loi dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » C'est donc en rejetant toute demande d'avantages spécifiques des associations cultuelles que l'État et les collectivités locales assurent le respect du principe de neutralité à l'égard de tous les citoyens et le libre exercice des cultes ou de l'absence de culte. Vous connaissez l'attachement viscéral de mon groupe à ces principes, qui se confondent avec notre République. C'est par conséquent dans le souci de les défendre qu'il s'oppose pour partie aux articles 25 et 38 du projet de loi de loi qui visent à faire bénéficier les associations cultuelles d'avantages pour compenser la diminution de leurs ressources, comme cela est expliqué dans l'exposé des motifs. Encore faudrait-il réaliser une véritable étude d'impact de cette question, qui est tout sauf anodine, vous et nous le savons bien.

Nous attendons, monsieur le secrétaire d'État, que vous ne l'éludiez pas. En conclusion, j'indique que, si mon groupe partage certains objectifs de ce projet de loi, notamment sur le droit à l'erreur et sur la philosophie qui le sous-tend, nous attachons une grande importance aux amendements relatifs à la loi de 1905 et au monde agricole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission spéciale, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi dont nous commençons l'examen est une étape importante dans l'histoire administrative de notre pays. Bien sûr, il y a déjà eu des textes relatifs aux relations entre l'administration et les citoyens, mais celui-ci me paraît revêtir une importance particulière. est important parce qu'il parle de la confiance. Certes, la confiance ne se décrète pas, elle ne se légifère pas, mais les conditions de transformation profonde de l'action publique peuvent- dans cet hémicycle, nous en sommes tous, me semble-t-il, convaincus -être infléchies. Ce que nous demandent ce texte et la disposition qui l'a, en quelque sorte, englouti, c'est de repenser la place de l'erreur dans la société française. L'erreur est humaine mais ne semble pas toujours française ; reconnaissons-le, la place pour le rebond est moindre dans ce pays qu'outre-Manche, outre-Atlantique ou en Asie. Beaucoup de décisions de vie sonnent encore comme des verdicts irrévocables, comme des choix définitifs et indélébiles. Jusqu'à récemment- admettons que ce soit encore un peu le cas -, notre pays s'est caractérisé par un cercle vicieux par prévention de l'erreur, par peur de l'échec, par crainte de la sanction, on tente moins, on entreprend moins, on risque moins. Le Léviathan, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le marché, c'est la somme terrible des projets reportés, enfouis ou abandonnés, dans un pays qui n'a pas toujours donné sa chance à la chance. Bien entendu, tout n'est pas justifiable ni pardonnable, mais posons quelques principes. Nous sommes tous faillibles, mais nous sommes souvent de bonne foi. On peut commettre une fois une erreur dans un domaine et se la faire expliquer par l'administration. Le droit à l'erreur cesse évidemment d'exister lorsqu'il devient un abonnement ou un réflexe, mais c'est un atout précieux que de se dire que l'on dispose de ce recours. Oui, chers collègues, tout le monde peut se tromper et c'est cette réalité que le présent texte souhaite rappeler.

Ce changement a évidemment des implications directes sur les relations entre l'administration et les administrés. Les attentes sont fortes, du côté que ce soit des usagers ou des agents publics. J'insiste sur ce point : les agents publics sont intimement attachés aux valeurs du service public, dont ils sont les garants, dont ils assurent la qualité.

concerne les usagers, le groupe La République en Marche rappelle son attachement à la pratique du rescrit, bien connu de l'administration fiscale ; un accord est souhaitable sur ce point. La simplification est presque devenue

Simplifier est une nécessité- je n'ai jamais rencontré d'de la procédure, de conservateurs de la norme, ni d'inconditionnels de la pièce manquante. C'est pourquoi je ne peux que me féliciter de voir des mesures de bon sens dans ce projet de loi ; c'est le cas du référent unique, mais également de l'interdiction faite aux administrations de recourir à des numéros surtaxés à l'horizon 2021. Comme La Fontaine avait affligé les animaux de la peste, notre pays est malade de la norme. Ce texte invite le législateur, c'est-à-dire le Gouvernement et nous, parlementaires, à stopper l'hémorragie normative, dont une partie provient de la surtransposition des textes de l'Union européenne. Ce projet de loi est aussi- peut-être d'abord -un texte qui fait du numérique un levier de transformation du service public. Cela est totalement cohérent avec les mutations profondes qu'internet implique et que le Gouvernement souhaite approfondir au travers de l'ambition de dématérialisation de 100 % des procédures. Internet constitue une transformation permanente, en raison de l'océan de données qui le traverse et qui est aussi un atout pour améliorer la qualité du service rendu. Nous devons encourager un État plateforme, aux méthodes plus agiles et au déploiement plus souple. Nous devons également utiliser le numérique comme un moyen d'évaluation des services publics par les usagers. C'est pourquoi le groupe La République en Marche a souhaité amender la stratégie nationale d'orientation de l'action publique en rendant disponibles les enquêtes internes de satisfaction de certaines administrations, en les anonymisant, évidemment. La confiance ne se décrète pas,

Le débat permettra par ailleurs d'éclaircir les recours aux ordonnances sur certains points. Sans abandonner notre mission d'évaluation, nous souscrivons à ce choix gouvernemental. Je tiens également à souligner l'importance de ce qui a été appelé le service après-vote, la nécessité pour les parlementaires de se soucier de l'application des différentes mesures contenues dans ce texte. Il faut que les mesures réglementaires soient prises pour faire en sorte que nos concitoyens perçoivent le changement de logique dans les têtes et dans les faits- c'est toute la philosophie du conseil de la réforme. Je conclus en indiquant que ce texte, loin d'affaiblir l'autorité de l'État, renforce celle-ci, en permettant aux citoyens, au travers de nouveaux droits, de casser ce que l'économiste Yann Algan a justement appelé la « fabrique cher collègue ! L'administration de demain, c'est davantage de liberté pour les usagers et davantage d'autonomie pour les agents, c'est un service public efficace et des lois mieux appliquées, car rendues plus applicables. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'ambition affichée par ce projet de loi est « de construire un État conscient de son coût, usant à bon escient de ses prérogatives, et oeuvrant tout entier à seconder la vie sociale et favoriser son épanouissement, un État au service d'une société de confiance. Ce texte traduit la vision d'un État « bienveillant et ouvert », selon l'exposé des motifs. Je ne reviendrai pas sur le titre même du texte, entre novlangue orwellienne et langage publicitaire ... selon une thématique et un discours déjà largement éprouvés depuis le début de la législature, il faudrait penser que l'État coûte trop cher et qu'il n'agit pas toujours comme il conviendrait. Pour remédier à cela, ce projet de loi hétéroclite et parfois difficile à appréhender dans ses conséquences concrètes prévoit simplement de codifier des pratiques administratives existantes ; loin de simplifier, il vise à cristalliser des pratiques administratives quotidiennes. De manière assez surprenante, il met en question en bien des domaines, singulièrement en matière de fiscalité des entreprises et des patrimoines, des pratiques qui attestent de longue date de la souplesse et de la flexibilité de l'administration devant l'examen des situations concrètes. Pour ne prendre qu'un seul exemple, parlons du droit à l'erreur, le produit promotionnel d'affichage du projet de loi, un droit qui n'a rien de nouveau et qui est pratiqué singulièrement en matière fiscale. En effet, le code général des impôts dispose à l'article 1729 que les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application » de

Quant à la transaction, elle est déjà fortement pratiquée, ne serait-ce que pour éviter qu'un contribuable indélicat, notamment une entreprise subissant un redressement, ne se retrouve dans la plus parfaite incapacité de payer.

De plus, tant le Conseil d'État que le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, ont signalé les risques d'atteinte au bon fonctionnement des administrations, dans le contexte budgétaire contraint qui leur est imposé depuis plusieurs années. En effet, ce texte doit être appréhendé dans le contexte actuel de mise en cause du statut des fonctionnaires, avec le « plan 2022 » de réduction d'effectifs et de développement des contrats de mission et autres emplois contractuels. Outre que la recette est passablement ancienne, comment peut-on faire de la bonne administration, avec la sécurité juridique et la confiance qui conviennent, quand on place les acteurs de cette administration en situation d'insécurité professionnelle ? Ainsi, le Conseil d'État estime que « ce dispositif, dont le champ d'application est extrêmement vaste, pourrait porter atteinte au bon fonctionnement de l'administration dès lors qu'il prévoit que celle-ci est tenue de faire droit à cette demande dans un délai raisonnable sans tenir suffisamment compte de ses moyens et de ses effectifs. Il relève que les moyens des services de l'État ont souvent été fortement réduits et ne lui permettent pas toujours d'assumer ses missions premières, au risque d'exposer la responsabilité de l'État et la responsabilité pénale de ses agents. » Non seulement ce projet de loi ne remet nullement en question les politiques qui, de révision générale des politiques publiques en modernisation de l'action publique, ont largement entamé la crédibilité du service public par l'abandon marqué de la présence territoriale des services déconcentrés des différentes administrations, mais encore il les prolonge et en accentue les défauts et travers, pour faire de cas d'espèce la matrice de la suraccumulation législative que nous connaissons. Sur un plan formel de légistique, observons que la majorité des articles du texte consiste en des habilitations à légiférer par ordonnance et en des dispositifs dérogatoires destinés à être expérimentés. Il prive ainsi la représentation nationale de bien des débats.

lui-même dans son avis « le risque de voir les dispositifs envisagés bénéficier essentiellement aux personnes déjà les plus à même de les mobiliser et de renforcer ainsi les inégalités d'accès aux droits ». Il est évident que, dans la société de confiance décrite par le texte, ce sera avocat-conseil pour les uns, et écrivain public pour les autres ... Enfin, la lutte contre la fraude fiscale et sociale, si chère à nos coeurs et priorité absolue des politiques publiques, semble curieusement curieusement absente de ce texte. Elle illustre pourtant par excellence la confiance des administrés envers l'État, dès lors qu'elle signe l'égalité de traitement, ainsi que la continuité du service public, en pleine et entière application du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. Là serait la véritable ambition de ce gouvernement : renforcer les systèmes déjà existants, donner les moyens aux agents d'assurer au mieux leur mission de service public. En effet, la relation de confiance entre l'administration et les usagers ne peut se créer que si le service public garde ses principes d'équité de traitement et de continuité. Cela, seul le statut actuel de la fonction publique le garantit. Ce n'est pas parce qu'il date de 1945 et qu'il a été rénové en 1984 qu'il ne recèle pas toute la modernité dont nous avons besoin en 2018 ! Améliorer la relation passe par une action publique renforcée sur le plan des moyens budgétaires autant qu'humains. Les garanties existent déjà pour les citoyens. Il faut donner aux agents du service public les moyens de les mettre en oeuvre, la proximité territoriale permettant à chaque citoyen d'être correctement informé de ses droits et obligations. Ce projet de loi, teinté d'une once de démagogie, n'est qu'une énième couche à l'indigeste millefeuille législatif qui a dévoyé le sens de l'action publique depuis une bonne vingtaine d'années. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission spéciale, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui pourrait se résumer en deux mots : « confiance » et « simplification ». Vous le savez autant que moi, la confiance ne se décrète pas. Elle s'obtient par l'action et par un travail quotidien. Une fois perdue, elle ne se regagne que difficilement. Or la trop grande complexité administrative et, pour ainsi dire, la déshumanisation des services publics auront, de proche en proche, contribué à dégrader la confiance des administrés dans leur administration. Il est ici question de la confiance réciproque entre citoyens et administration, mais également de la confiance des entreprises en l'efficacité de l'État. Ce projet de loi procède du constat selon lequel l'imbrication des procédures entrave trop souvent le bon fonctionnement des services publics, alimentant à mesure la défiance des particuliers comme des entreprises. Afin de simplifier les procédures auxquelles, chaque jour, des millions de Français sont soumis, afin de restaurer le lien de confiance qui doit unir chacun d'entre nous à l'administration, nous devons préférer l'action aux propos incantatoires. Tel est l'objet de ce texte. Il faut s'en féliciter. Cependant, avec ce projet de loi, il s'agit de regrouper la totalité des mesures de simplification voulues par le Gouvernement que d'améliorer l'ensemble des procédures, des recours et des relations entre l'administration et le public. On ne peut qu'être d'accord avec cet objectif. Aussi saluerai-je la sagacité de la commission spéciale et de ses rapporteurs, qui ont su veiller à la qualité législative, en évitant de transformer ce texte en une loi fourre-tout, tout en lui ôtant ses mesures jugées superfétatoires. Dans sa version transmise par l'Assemblée nationale, le projet de loi prévoyait, en effet, un grand nombre de rapports, pas toujours utiles- les membres du Parlement en savent quelque chose -, et habilitait de manière démesurée le Gouvernement à réformer par voie d'ordonnance. Je prendrai, à ce titre, l'exemple de l'article 26, qui a été très justement supprimé par la commission, car il retirait au législateur ses compétences en matière de création et de fonctionnement des modes d'accueil de la petite enfance. La commission a, ainsi, veillé au respect des compétences du Parlement. Ce ne peut être qu'une bonne chose mes chers collègues, de revenir sur quelques mesures symboliques du projet de loi. Je le ferai en trois points. Il s'agit, tout d'abord, de la confiance de l'État en la bonne foi des citoyens. L'article 2 symbolise, en ce sens, l'esprit et la philosophie du texte. Le droit Le droit à l'erreur qu'il introduit va permettre une certaine réhumanisation des rapports entre citoyens et administration. Tout le monde peut se tromper en étant de bonne foi. C'est pourquoi il nous semble primordial qu'avant toute sanction l'administration puisse, dans un périmètre nécessairement délimité, inviter l'usager à régulariser sa situation. ce qui est de l'instauration du droit au contrôle opposable, en fixant un délai maximal de six mois, la commission spéciale l'a rendu effectivement opérationnel et véritablement incitatif. De même, un citoyen de bonne foi ne perdra plus le bénéfice d'un avantage fiscal s'il manque à une obligation déclarative. Il bénéficiera aussi de l'intervention d'un médiateur en cas de conflit avec les organismes de sécurité sociale. Il s'agit, ensuite, de la confiance réciproque- et nécessaire ! -entre l'État et les collectivités territoriales. À propos du chapitre I, nous devons, en tant que représentants des collectivités territoriales, nous réjouir de l'article 2 A, introduit lors des travaux de la commission, sur l'initiative de notre collègue Sylvie Vermeillet, qui étend aux collectivités le droit à régularisation en cas d'erreur. Par ce biais, les relations que les collectivités entretiennent avec l'État ou avec les organismes de sécurité sociale s'en trouveront apaisées, la bienveillance de l'État envers elles induisant une reconnaissance de leurs mérites dans la conduite de missions parfois difficiles à accomplir. Il s'agit, enfin, de la confiance mutuelle entre l'État et les entreprises. comme les citoyens et les collectivités, les entreprises ont elles aussi besoin d'avoir confiance dans l'État pour prospérer et faire avancer le pays. Ainsi, l'article 7, qui donne la priorité à l'accompagnement continu des entreprises dans leurs obligations déclaratives et qui inscrit dans la loi le souhait qu'avaient émis bon nombre d'entre elles, va dans le sens d'une relation de confiance. De même, la durée des contrôles administratifs sur les TPE et les PME sera limitée. Ce sont là des mesures que nous approuvons. L'administration est, bien entendu, au coeur même de ce texte. Sans elle, aucune confiance n'est possible. Sans elle, il n'y a pas de lien avec les citoyens et, en définitive, pas de services publics ! C'est pourquoi il est indispensable que le Gouvernement alloue effectivement à la formation des fonctionnaires la somme de 1,5 milliard d'euros prévue sur les cinq prochaines années. Ce n'est que par les fonctionnaires que la réforme deviendra effective. Il est, par exemple, impensable que l'administration puisse, avec la création puis l'extension du certificat d'information prévues à l'article 12, répondre dans les trois mois à l'usager sans ces moyens nouveaux. Mais, malgré ces quelques mesures satisfaisantes, nous ne devons et ne pouvons pas nous contenter de ce projet de loi. Le travail n'est pas fini. Ce texte est un premier pas, pas, utile, mais insuffisant. Je le répète : la confiance est quelque chose qui se construit. Et, comme pour toute construction, il faut que les bases soient solides. C'est pourquoi, tout comme nous serons vigilants lors de la ratification des ordonnances, nous veillerons à ce que les décrets d'application soient bien pris et à ce que les expérimentations fassent l'objet d'évaluations. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous sommes favorables à ce texte et aux idées qui le sous-tendent. Si l'ambition est grande, il faudra cependant redoubler d'efforts

Les conditions d'examen du texte ont été marquées par deux particularités. Tout d'abord, nous avons constitué une commission spéciale, réunissant des parlementaires de différentes commissions. Les sept commissions permanentes étaient représentées. Certes, le choix de la commission spéciale soulève encore des réticences quand plusieurs commissions s'estiment compétentes sur un même texte. Au vu de notre expérience, je crois pouvoir dire cependant que cette formule a été appréciée, parce qu'elle permet de réfléchir ensemble, dans la diversité de nos compétences, et de nous enrichir mutuellement de nos expériences respectives. La commission spéciale a également eu l'honneur de mettre en application, pour la première fois, la procédure de législation en commission, telle qu'elle résulte de la modification de notre règlement en date du 14 décembre 2017, plus précisément sa nouvelle formule, qui est la législation partielle en commission. Nous avons montré, je crois, que cette procédure n'enlevait rien à la qualité des débats ni au sérieux de l'examen des dispositions d'un projet de loi.

procédure est particulièrement bien adaptée aux textes techniques, les débats sur les politiques lourdes ayant évidemment vocation à demeurer effectués en séance publique, selon la procédure classique. Pour un bon usage de la législation en commission, il est aussi important de conclure un pacte de confiance entre les parlementaires des différentes sensibilités compte tenu des différentes possibilités d'utilisation du veto qui sont aujourd'hui inscrites dans les textes. Dans le cas de la législation en commission partielle, le choix des articles est évidemment essentiel. La principale difficulté réside dans les délais très courts qui nous sont donnés pour effectuer ce tri et présenter des propositions satisfaisantes. état de cause, cette première expérience montre que le Sénat sait moderniser et simplifier son mode de fonctionnement, privilégiant la fluidité et l'efficacité au service de la qualité dans l'élaboration de la loi. Je dois reconnaître, sur cet aspect de procédure législative, un contraste certain avec les manières du Gouvernement, qui sont à l'opposé de relations de confiance avec le Parlement,

La commission spéciale a cherché à recueillir le plus d'observations et d'avis possibles sur les différentes mesures qui figurent dans le projet de loi, d'abord par le biais des auditions tenues en réunion plénière, mais aussi

La commission a également recueilli sur internet les contributions de nos concitoyens, acteurs publics ou usagers des services, un espace participatif que nous avons ouvert. Nous avons été très intéressés par ces contributions, de grande qualité, dont une sélection figure d'ailleurs en annexe au rapport de la commission. À titre personnel, j'ai aussi organisé des réunions avec les services déconcentrés de l'État, en particulier la direction départementale des finances publiques, la direction départementale des territoires, le préfet et ses services, mais également les élus locaux, maires et présidents d'intercommunalité.

mais, assez rapidement, on passe à la perplexité, si ce n'est à la déception. Le sujet que nous abordons au travers de ce projet de loi, celui des relations entre le public et les administrations, soulève, en effet, beaucoup d'attentes nos concitoyens- particuliers, associations et entreprises -demandent plus de simplicité, plus de bienveillance et de souplesse, plus de rapidité dans le traitement des demandes, plus d'attention et de conseil. Au reste, ces demandes légitimes se renforcent face à deux phénomènes un droit qui se complexifie et une société qui s'habitue à des réactions rapides, voire immédiates, du fait des technologies numériques- on pose une question et on veut une réponse dans la seconde. L'intitulé du projet de loi et son annexe renvoient ainsi à une société où tout est réglé en deux clics, où le citoyen-contribuable-usager gère ses situations administratives internet, dont il maîtrise évidemment toutes les subtilités, et où l'erreur qu'il peut commettre est aussitôt corrigée par une administration disponible et indulgente. C'est merveilleux ! Cette vision idéalisée est pourtant contredite par certaines réalités, et d'abord par les inégalités dans l'accès aux procédures dématérialisées, soit pour des raisons d'infrastructures défaillantes dans nos territoires, soit pour des raisons culturelles et sociales. Pensons à ceux que l'on appelle les « invisibles », les « illettrés » du numérique. En légiférant, nous devons toujours avoir présent à l'esprit le caractère universel de la portée de la loi.

de l'administration ne sont pas à la hauteur. Je pense tout particulièrement à l'archaïsme des systèmes d'information de l'État et de leurs applications logicielles.

trop souvent constaté entre les ambitions déclarées et les moyens que vous nous donnez. L'histoire récente des relations entre l'administration et les citoyens est malheureusement est malheureusement celle d'une succession de lancements de démarches-qualité sans évaluation des résultats, de plans de communication mal suivis d'effets. Ce n'est pas ainsi que l'on renforce la confiance. Il est à craindre que ce texte ne s'inscrive dans cette lignée. Vous souhaitez faire passer l'action publique d'une logique de moyens à une logique de résultat. Nous partageons l'objectif. C'est un bouleversement considérable. Veuillez conclure, mon cher collègue.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission spéciale, madame la rapporteur, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Jérôme Durain l'a rappelé tout à l'heure, ce texte de loi pour un État au service d'une société de confiance nous a permis d'aborder une multitude de sujets tenant aux relations entre les citoyens, les entreprises et l'administration. C'est un exercice particulier pour notre assemblée, peu habituée à débattre, dans ce format et sur un même texte, de sujets aussi divers que le rescrit fiscal, le code des douanes, le droit du travail, le régime d'autorisations environnementales ... J'en passe. Cette accumulation nous a inquiétés, ne nous en cachons pas. Nous n'avons pas toujours perçu de quelle manière cet amoncellement de sujets aussi variés et abordés de façon parcellaire pouvait créer les conditions d'une société de confiance. Patchwork d'idées, réécriture législative de dispositions récemment adoptées : sur la méthode de travail, la confiance n'était pas toujours au rendez-vous. sur l'ambition de simplification, ce projet de loi me semble passer à côté de l'enjeu essentiel : s'assurer que l'administration est toujours présente, effective, pour accompagner les plus fragiles. En matière de patchwork, j'avais fait part, en commission spéciale, de mon très grand étonnement à la lecture de l'amendement gouvernemental visant à instaurer l'article 26 relatif à l'habilitation à prendre, par ordonnances, toute toute mesure facilitant l'implantation, le développement et le maintien de modes d'accueil de la petite enfance. Ces dispositions, en vigueur dans plusieurs types d'établissements- crèches, microcrèches, multi-accueils qui diffèrent par leurs statuts et leurs modes de gestion- associative, municipale ou intercommunale, publique ou privée -, méritent un plus large débat que celui que permet une simple ordonnance. Il s'agit de la vie quotidienne de près de 900 000 enfants accueillis, de leurs parents

très récents de notre législation, tout juste entrés en application, sans attendre que l'encre sèche. Instaurer une société de confiance mérite de prendre le temps et le recul nécessaire pour évaluer les dispositions en vigueur À cet égard, l'article 33 relatif à la simplification des modalités de consultation du public lors de la création d'installations classées pour la protection de l'environnement venait heurter de plein fouet de très récentes dispositions. Je me félicite également que seule la consultation électronique ait été supprimée et que le Sénat ait donc choisi de renforcer l'évaluation de la participation du public. La méfiance suscitée chez nos concitoyens par certaines installations agricoles intensives, par exemple, nécessite que l'on conserve des procédures de consultation humanisées, en présence des commissaires enquêteurs. Plus d'humanité, plus d'attention à l'égard de nos concitoyens les plus fragiles, c'est ce qui devrait caractériser une administration soucieuse d'instaurer un climat de confiance. Pourtant, ce n'est pas à ce défi que s'attaque ce projet de loi. Nous le regrettons. Sur le plan des moyens humains accordés à l'administration publique, le compte n'y est pas, comme mon collègue l'a rappelé. Sur un autre plan, votre projet de loi, monsieur le secrétaire d'État, manque d'ambition : il ne répond aucunement à l'exigence d'un réel accès aux droits.

Avec mes collègues socialistes, j'espère que cet examen en séance aboutira à la mise en place d'un dispositif ambitieux qui consacre une part des économies réalisées par la dématérialisation de notre administration au profit de la réduction de la fracture numérique. Nous ne pouvons nous résigner à ce que nombre de nos concitoyens se voient rejeter d'un système de plus en plus déshumanisé, robotisé, où l'algorithme décide et exclut les illettrés numériques. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, faute d'y voir un acte majeur de simplification administrative et une remise au premier plan d'une administration inclusive, nous nous abstiendrons sur ce texte.

la délégation sénatoriale aux entreprises- j'ai l'honneur de présider celle-ci -ne font pas un seul déplacement sur le terrain sans entendre les entreprises déplorer la complexité de l'administration et dénoncer son approche sourcilleuse, voire suspicieuse.

à orienter l'administration vers le service aux entreprises, notamment en donnant la priorité à la simplification », et à « passer d'une logique reposant sur la défiance [ ...] à une logique fondée sur la confiance. Vous le voyez, le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui s'inspire largement des travaux de notre délégation. Nous ne pouvons que nous en féliciter. La stratégie nationale d'orientation de l'action publique vers une société de confiance, annexée à l'article 1, nous brosse le tableau d'un monde idéal, où l'administration facilitera enfin la vie des entreprises et leur fera confiance. Nous rêvons, avec vous, monsieur le secrétaire d'État, que l'impulsion que veut donner ce texte soit suivie d'effets concrets. Mais notre rêve ne va-t-il pas tourner court ? Par exemple, la prise en compte de la capacité financière du contribuable, proclamée dans cette annexe, ne trouve pas dans le texte de déclinaison concrète pour les entreprises. De même, l'objectif de simplification affiché ne va pas assez loin : il faudrait s'assurer que la création d'une norme nouvelle entraînant une charge supplémentaire pour les entreprises s'accompagne de l'abrogation de normes représentant une charge au moins équivalente. La délégation aux entreprises accompagne donc le changement d'état d'esprit que marque le texte, mais elle est lucide sur le caractère largement incantatoire de l'ensemble de ses dispositions. Diverses mesures, apparemment séduisantes, sont décevantes à l'examen prévoir que l'absence d'une pièce non essentielle dans un dossier ne peut pas conduire l'administration à suspendre l'examen de la demande, c'est bien, mais savoir pourquoi cette pièce est demandée par l'administration, alors qu'elle n'est pas essentielle, serait tout de même beaucoup mieux ! Consacrer la procédure du rescrit contrôle est sans doute utile, mais simplifier le code général des impôts le serait bien davantage. Et les rares surtranspositions sur lesquelles le texte revient, en matière environnementale, ont été introduites par ordonnances en août 2016 et janvier 2017. L'important est donc de trouver comment discipliner l'administration, plutôt que de rectifier après coup, ce qui nourrit l'instabilité législative. En outre, de nombreuses avancées prévues par le texte sont soumises à des exclusions, des conditions ou des expérimentations qui en réduisent considérablement la portée. Ainsi, pour mettre en oeuvre le principe « dites-le-nous une fois », votre texte ne propose qu'une expérimentation sur quatre ans et renvoie à un décret en Conseil d'État la délimitation du champ des données concernées. Or ce sont 10,7 millions de pièces justificatives que l'administration sollicite chaque année. La simplification est donc urgente. L'expérimentation, réduite, est-elle à la hauteur de l'enjeu ? Au total, la volonté du Gouvernement de faciliter la vie des entreprises apparaît bien timide. Aussi, nous vous proposons d'aller plus loin, en soumettant l'administration à une évaluation régulière par les entreprises et en se donnant les moyens de simplifier le droit applicable aux entreprises. En Allemagne, le, le NKR, a permis d'alléger la charge administrative de 14 milliards d'euros en cinq ans. C'est pourquoi nous pensons que le plus efficace serait de charger un organe d'améliorer le droit pour les entreprises et de procéder à la contre-expertise des études d'impact produites par l'administration.

Monsieur le secrétaire d'État, il est difficile d'identifier la portée réelle des textes que le Gouvernement nous présente, au-delà du vocabulaire employé et de la communication devenue habituelle. Ainsi, ce projet de loi a été présenté par le ministre de l'action et des comptes publics comme une révolution des relations entre l'administration et les Français. Or, comme souvent, le champ de la révolution annoncée est bien moins important que la communication qui en a été faite.

Nombre d'amendements déposés en commission spéciale ont été rejetés comme étant des cavaliers législatifs. J'espère vivement que les amendements de séance déposés, visant en particulier à lutter contre les surtranspositions dans le secteur agricole, où elles sont si incomprises,

les majorations de 40 % ou de 80 % ne peuvent être appliquées que si l'administration apporte la preuve d'une intention de frauder. En matière douanière, les infractions font l'objet d'une transaction dans 99 % des cas, aboutissant, pour 20 % d'entre eux, à la suppression totale des pénalités.

L'autre disposition substantielle du texte concerne la généralisation de la relation de confiance, inscrite à l'article 7. Expérimentée depuis 2013, elle consiste à valider en amont les options fiscales d'une entreprise dans le cadre d'un dialogue et sur une base contractuelle. Il s'agit d'une avancée dont

sollicitation. Le texte prévoit, à l'article 16, d'expérimenter, dans deux régions, une limitation de la durée cumulée des contrôles administratifs sur les PME. Toutefois, ce principe est déjà assorti de nombreuses exceptions.

à la suite de la publication d'un rapport sur l'accueil à distance dans les administrations sur le site internet de l'Inspection générale des finances, enjoint les centres d'appels des principales administrations à facturer leurs appels au prix d'une communication locale. Il faut malheureusement en déduire que les consignes données par un gouvernement sont encore loin d'être respectées par nos administrations. C'est dire s'il y a lieu de modifier la culture et les habitudes d'un certain nombre d'entre elles.

de ce même grand plan d'investissement d'avenir, un fonds de 700 millions d'euros sur cinq ans consacré à la modernisation des administrations. Nous partons du principe que, pour se moderniser, pour être plus efficace, il faut savoir payer et doter nos administrations de nouveaux outils.

accepter en l'état l'article 1 de ce projet de loi et le contenu de son annexe reviendrait à renoncer, par principe, aux vertus fondatrices du service public à la française. Dans les faits, au-delà des apparences nécessaires d'une relation courtoise et humaine entre administrés et administration, c'est bel et bien la capacité du service public à agir avec des effectifs de plus en plus réduits- la programmation de 120 000 suppressions de postes, que vous assumez, monsieur le secrétaire d'État, demeurant inscrite à l'arrière-plan du débat question. L'administration de conseil et de service que semble vouloir promouvoir ce projet de loi nous apparaît comme une réponse malthusienne de réduction des services humains, remplacés par des procédures toujours plus automatisées. C'est non pas l'accumulation des services et leur organisation qui pose parfois problème aux administrés, mais bien plutôt les pressions contradictoires exercées à leur endroit. Prenons l'exemple des administrations fiscales : ces dernières sont mises en demeure, depuis le vote de la loi de finances rectificative pour 2012, de promouvoir auprès des entreprises le crédit d'impôt pour la compétitivité et et l'emploi tout en luttant contre la fraude fiscale. Or une activité de contrôle fiscal n'est pas qu'affaire de « gros coups », mais constitue plutôt une activité unissant les services fiscaux, du plus obscur des centres de finances publiques jusqu'aux directions spécialisées les plus pointues, pour faire respecter le principe d'égalité devant l'impôt, principe fondateur de nos valeurs républicaines. Nous faisons nôtres les préoccupations du Conseil d'État : ajouter aux procédures de l'administration l'exercice du droit au contrôle par le contribuable ou par l'administré en général risque fort de poser des problèmes d'organisation. Ce phénomène a été relevé plusieurs fois par les syndicalistes des finances sur le contrôle fiscal. Le contrôle fiscal externe a toujours été considéré par les pouvoirs publics comme une vitrine de l'action de l'administration fiscale et de la lutte contre la fraude, une vitrine que chaque ministre et directeur général s'échinent à lustrer, alors qu'il y a de moins en moins de choses en magasin.

Il nous a d'abord paru indispensable de rappeler que les services publics ont pour vocation essentielle de répondre aux besoins de la collectivité, c'est-à-dire aux attentes de la population dans la diversité des situations. N'oublions pas que ce lien s'est pour le moins distendu du fait notamment de politiques publiques ayant tourné le dos aux fondamentaux du service public- égalité, continuité, neutralité, accessibilité et laïcité -pour mener des politiques sélectives s'éloignant toujours un peu plus de la justice sociale la plus élémentaire. Il est évident qu'une véritable action publique ne peut avoir de pertinence et de résultats qu'en s'appuyant pleinement sur ses propres ressources humaines, source de la valeur ajoutée, portée par l'action publique au bénéfice de l'ensemble de la collectivité. Le statut de la fonction publique recèle un puissant potentiel de mise en mouvement des agents publics et tend notamment à valoriser et leurs compétences et leur qualification. Dans l'absolu, la formation continue des agents publics ne peut se contenter d'une simple adaptation de ces agents à je ne sais quelle nouvelle technologie ou quelle bonne pratique sans reconnaissance quelconque de cette évolution. De fait, la fonction publique est un ensemble de métiers tout à fait exceptionnels, loin de l'image courtelinesque des ronds-de-cuir, faits de savoirs, de savoir-faire, de gestes professionnels qu'il convient de valoriser et dont la pleine expression est l'un des enjeux à venir. La lecture de l'article 29 du présent projet de loi suffit à montrer, si besoin était, que l'on ne peut se contenter d'expédients et de solutions à l'emporte-pièce en la matière et qu'il est grand temps d'envisager la question sous tous ses aspects systémiques la place des personnes âgées dans notre société, par exemple ; la qualité des services que nous pouvons apporter ; le statut ; les compétences et la reconnaissance que nous pouvons accorder à ceux dont le métier est, ou sera, demain, d'assister ; les sommes que nous sommes disposés à consacrer à la satisfaction de ces besoins ... Voilà, selon nous, quel est l'enjeu et comment donner du sens

Cet amendement vise à insérer dans la stratégie nationale d'orientation de l'action publique un alinéa aux termes duquel « l'application par l'administration des principes et droits au bénéfice des usagers est conditionnée à une exigence de respect et de courtoisie des usagers envers l'administration. » Évident, me dira-ton, mais cela va

parole est à M. le secrétaire d'État. Cet amendement vise à introduire dans la stratégie nationale une nouvelle orientation selon laquelle toute personne a accès à une information transparente sur l'efficacité et la qualité du service public en relation avec les usagers.

Selon l'OCDE, cette complexité administrative coûte chaque année 60 milliards d'euros à l'économie française. Nos entreprises souffrent de ces charges administratives, fiscales et sociales particulièrement lourdes qui nuisent à leur compétitivité. Le législateur doit en tenir compte et accepter comme objectifs contraignants la simplification des normes et la stabilisation, voire l'allégement, des charges applicables aux entreprises. Les auteurs de cet amendement proposent donc que les normes supprimées

Qu'il s'agisse de personnes résidant dans des zones blanches, de personnes non dotées de matériel informatique ou de personnes ne maîtrisant pas l'outil numérique, ces dernières se retrouvent dans l'incapacité d'effectuer les démarches requises.

Le ministère de l'économie et des finances annonce une économie de plus de 60 millions d'euros, liée à la dématérialisation des feuilles d'impôts, des passeports, des permis de conduire ... Il serait souhaitable qu'une partie de ces économies réalisées par la baisse des coûts soit prioritairement mobilisée pour la mise en oeuvre de mécanismes d'accompagnement des publics exposés au risque de marginalisation numérique. En effet, dans la mesure où ce projet de loi vise à la fois à la dématérialisation de nos services publics et à une simplification de l'accès aux informations par les usagers, il ne saurait créer un mécanisme de renforcement des inégalités territoriales et sociales. Refonder les relations public-administration ne revient pas à exclure encore davantage. L'adoption de cet amendement devrait permettre de renforcer l'accès au droit. Voyez-le comme une clause de protection des publics vulnérables.

Je veux excuser l'absence de M. le Premier ministre, qui m'a téléphoné : il est retenu à l'Assemblée nationale par l'examen du projet de loi organique relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.

Suivre des formations professionnelles tout au long de sa vie apparaît aujourd'hui comme une nécessité incontournable. Les métiers changent ; les emplois se transforment ; nous devons tous nous adapter. Cette adaptation s'inscrit dans le temps. Elle n'est plus ponctuelle comme elle le fut autrefois ; elle est continue et permanente. Il nous appartient, en tant qu'hommes et femmes du XXI siècle, d'accompagner ce changement. À titre individuel, chacun d'entre nous doit fournir cet effort de remise en question des connaissances acquises, pour choisir la ou les bonnes formations du futur. C'est pourquoi nous parlons désormais d'un parcours de formations au pluriel, à réaliser tout au long de notre carrière. Votre réforme, madame la ministre, est innovante. Elle place le salarié au coeur du dispositif : il a la liberté de choisir son avenir professionnel. Elle ne néglige pas pour autant l'entreprise, puisque celle-ci peut proposer et organiser des plans de formations spécifiques à son activité. Elle protège les salariés les plus vulnérables. Par exemple, elle attribue une somme forfaitaire à chacun des salariés, quelles que soient la rémunération et la taille de l'entreprise qui l'emploie. Alors que les partenaires sociaux avaient trouvé un accord très positif et très constructif, vous n'avez pas hésité, avec un courage certain, à aller au-delà de cet accord.

madame la ministre, de bien vouloir expliciter les motifs qui vous ont amenée à adopter ce nouveau système de décompte qui peut apparaître pour les uns comme un pari risqué et pour les autres comme une avancée majeure. La parole

notre système de formation professionnelle, qui avait de l'avance voilà trente ans, ne répond plus aux enjeux des grandes mutations technologiques, économiques et écologiques qui s'annoncent. Il est aussi inégal et injuste. Aujourd'hui, un ouvrier ou un employé a deux fois moins de chances qu'un cadre de se former. Et ce ne sont pas les cadres qui se forment trop ! La raison tient à ce que nous n'investissons pas assez dans la qualification des ouvriers et des employés. Un salarié d'une PME a deux fois moins de chances de se former

! Demain, il sera beaucoup plus facile de trouver une formation, de la comparer en ligne, de connaître les taux d'insertion et les taux d'accès au diplôme, de s'enregistrer et de payer directement. C'est également beaucoup plus juste.

La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Du 19 au 21 mars prochains, le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg seront en visite en France, sur invitation du Président de la République. Cela fait près de quarante ans qu'une telle visite n'avait pas eu lieu. En marge de celle-ci, M. le Premier ministre et son homologue luxembourgeois présideront un séminaire intergouvernemental. C'est sur les enjeux transfrontaliers que je souhaite attirer l'attention Être voisin du Luxembourg est le plus souvent une opportunité : 90 000 Français y travaillent et la dynamique économique se poursuit. En conséquence, 12 000 voyageurs empruntent quotidiennement la ligne TER Nancy-Luxembourg et 100 000 véhicules circulent sur l'autoroute A31. Ces chiffres sont en constante augmentation. Cependant, les enjeux transfrontaliers dépassent cette seule question de la mobilité. La compétitivité fiscale et sociale du Luxembourg pénalise le développement économique du côté français, bon nombre d'entreprises privilégiant leur installation au Luxembourg. Quant aux salaires, ils y sont de 30 % à 50 % supérieurs. Cette attractivité a de fortes répercussions, notamment auprès des professionnels de santé, lesquels, une fois formés, vont en grande partie exercer leur métier au Luxembourg, aggravant nos difficultés d'accès aux soins. Les défis à relever sont considérables pour corriger les effets d'un tel différentiel. Une mise en commun des moyens de la France et du Luxembourg, avec le concours de la région Grand Est, sur des projets coconstruits permettrait de répondre aux enjeux majeurs qui touchent directement la vie quotidienne des milliers de citoyens dont je me fais aujourd'hui la porte-parole. Comme le confirme le rapport du CGET, le Commissariat général à l'égalité des territoires, la multiplicité des acteurs du côté français et le morcellement de la gouvernance des territoires sont des freins supplémentaires à la reconversion du Nord lorrain. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous éclairer sur les propositions du Gouvernement pour contribuer au développement harmonieux de cette zone transfrontalière, où les espoirs sont immenses ?

vous avez raison de souligner le caractère exceptionnel de la venue du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse de Luxembourg à Paris. Cela n'était pas arrivé depuis 1978

Vous l'avez souligné, la dynamique transfrontalière est porteuse d'opportunités, mais aussi de défis, auxquels le séminaire susvisé contribuera à répondre. Nous souhaitons tout particulièrement évoquer avec le Luxembourg la facilitation de la vie quotidienne des 90 000 travailleurs frontaliers, en prenant des engagements communs, afin de cofinancer des infrastructures à leur bénéfice. Je pense tout particulièrement aux infrastructures de transport. Cela fera partie des discussions que nous aurons sur le rééquilibrage de la relation transfrontalière, y compris, madame la sénatrice, avec l'objectif d'un retour de l'impôt sur le revenu que le Luxembourg prélève sur nos frontaliers. Enfin, plusieurs accords de coopération bilatérale viseront à répondre aux difficultés concrètes que vous venez de souligner. Nous travaillons notamment sur des mesures dans le domaine de l'apprentissage, de la formation et de l'enseignement supérieur. Si je ne peux pas vous donner, madame la sénatrice, les conclusions de ce séminaire avant qu'il n'ait eu lieu, je peux vous affirmer qu'il se présente sous les meilleurs auspices.

au terme de cinquante jours d'offensives et de crimes commis en territoire syrien contre le peuple kurde, l'armée turque a déclenché depuis samedi un bombardement intensif de la ville d'Afrine. Au sol, les troupes turques et les forces de Daech repoussées vers le nord de la Syrie convergent pour faire tomber la ville. Tous s'apprêtent à commettre une tuerie irréparable, un massacre contre la population d'Afrine et les civils innocents qui y vivent.

Erdogan vise aussi à Afrine la remise sur pied d'une nouvelle base arrière de groupes criminels djihadistes, pour qu'ils reprennent leurs agissements terroristes. Les peuples kurdes et ceux de la région, comme nous-mêmes, en paieraient de nouveau le prix très cher. La cause des Kurdes est donc une nouvelle fois la nôtre. Il y a urgence à stopper Erdogan. C'est une affaire d'heures et de jours. La France doit réagir énergiquement et cesser ses ambiguïtés, au nom de l'appartenance de la Turquie à l'OTAN

pour interdire le survol d'Afrine par l'aviation turque et exiger que les troupes d'Ankara quittent la Syrie ? Il est encore temps d'arrêter la folie meurtrière d'Erdogan et de sauver Afrine. Nous demandons au Gouvernement d'agir, et d'agir vite.

l'opération que conduit la Turquie depuis maintenant cinquante jours dans le canton d'Afrine atteint un stade grave et critique, vous l'avez souligné. Plusieurs centaines de milliers de civils, dont beaucoup sont déjà des déplacés, attendent, privés d'eau et d'électricité, un assaut que les Turcs présentent comme imminent. Cela signifie des combats de rue, dont les populations paieront inévitablement le prix. Je voudrais faire quatre remarques Premièrement, le souci de protection des frontières, aussi légitime soit-il, ne peut en aucun cas justifier des opérations militaires aboutissant à des actions contre une population civile. Deuxièmement, la lutte contre Daech est la première raison de notre engagement militaire au Levant, et c'est une priorité de sécurité nationale.

L'armée turque a coupé l'alimentation en eau et en électricité de la ville d'Afrine, qui abriterait 800 000 personnes. Cette population assiégée, qui manquait déjà de médicaments et de vivres, est aujourd'hui en grand danger. Je veux rappeler en cet instant que les Kurdes ont été et sont nos plus précieux alliés dans la guerre contre les djihadistes. En leur infligeant une défaite cinglante à Kobané en 2015, en participant à la libération des territoires syriens aux mains de Daech, les Kurdes ont sacrifié leurs vies pour notre liberté. Ils ont eu un rôle déterminant aux côtés de la coalition.

pour arrêter cette violation du droit international par la Turquie, pour éviter les massacres de grande ampleur qui s'annoncent et pour empêcher que les Kurdes syriens soient aujourd'hui sacrifiés

Je me suis rendu à Moscou et à Téhéran voilà peu de jours pour dire, au nom du Président de la République, à mes interlocuteurs, au plus haut niveau, la manière dont la France concevait la situation en Syrie.

permettant l'acheminement de l'aide humanitaire et ouvrant la possibilité aux populations les plus touchées de regagner un lieu hospitalier

il ne s'est pas passé une seule journée sans que cette résolution ait été violée par le régime, qui a poursuivi ses offensives et ses bombardements contre les zones habitées. zones habitées. Des centaines de civils, qui attendent des soins médicaux d'urgence souvent vitaux, n'ont pas pu être évacuées ; les médicaments sont retirés des convois humanitaires.

la position de la France, c'est de faire en sorte que le droit international soit respecté. La France choisit le droit international plutôt que la guerre. C'est son objectif permanent, et elle le défend auprès de tous ses interlocuteurs.

En Europe, nous avons la même, mais en vrai. Et notre Franck Underwood s'appelle Martin Selmayr. M. Selmayr vient d'être nommé secrétaire général, le plus haut poste de la Commission européenne. Le seul problème, c'est qu'il n'en avait pas le droit. Le règlement est clair : pour devenir secrétaire général, il faut avoir occupé un poste de directeur. Or tel n'était pas le cas de M. Selmayr. Qu'à cela ne tienne ! Le 21 février dernier, sans les avoir prévenus de quoi que ce soit, Jean-Claude Juncker propose aux commissaires européens la nomination de Martin Selmayr au poste de secrétaire général adjoint. Puis il leur indique- heureuse coïncidence ! -que le secrétaire général, Alexander Italianer, vient de démissionner et que, en conséquence, il nomme M. Selmayr secrétaire général, poste qu'il a désormais le droit d'occuper puisqu'il est depuis neuf minutes secrétaire général adjoint J'ajoute qu'un appel à candidatures pour le poste de secrétaire général adjoint, obligatoire, mais réalisé de façon particulièrement discrète, n'avait suscité que deux réponses, celle de M. Selmayr et celle de sa collaboratrice, Clara Martinez. Dès la clôture des candidatures, personne ne pouvant plus candidater, Mme Clara Martinez retirait la sienne. Dans la foulée, le poste de chef de cabinet étant désormais vacant, Clara Martinez était nommée chef de cabinet. Ce coup de force illégal pose au moins deux problèmes. Le premier, c'est que, à un an des élections européennes, on ne peut faire plus grand cadeau aux europhobes, qui vont pouvoir dénoncer l'opacité, les manoeuvres internes, le manque de démocratie qu'ils reprochent à l'Europe. Le deuxième, c'est que désormais trois des principales directions européennes sur quatre sont tenues par un Allemand, déséquilibre contraire à toutes les traditions de partage des responsabilités entre pays membres. Le Parlement européen a convoqué hier une session en urgence qui a été houleuse et au cours de laquelle une enquête a été décidée. Mais le silence du Conseil européen, qui représente les gouvernements européens, est assourdissant. Ma question est simple, monsieur le ministre : comment la France compte-t-elle réagir à ce coup de force ? M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. sénateur Claude Malhuret, les nominations à des postes d'encadrement supérieur de la Commission européenne, tels que celui de secrétaire général, relèvent de la compétence stricte de la Commission, conformément aux textes en vigueur. Ces nominations sont décidées par le collège des commissaires. Il revient dès lors à la Commission d'apporter le cas échéant des précisions sur la procédure administrative suivie pour la nomination du nouveau secrétaire général. Le commissaire Oettinger était lundi devant le Parlement européen pour expliquer les raisons pour lesquelles la Commission considère que les règles en vigueur ont été respectées. La procédure se poursuit au Parlement européen. La France, qui n'est pas formellement impliquée, comme d'ailleurs les autres États européens, considère que les considère que les recrutements et promotions au sein des institutions européennes doivent répondre à des critères de mérite, de transparence, d'égalité des chances et d'équilibre géographique.

Les gouvernements Ayrault et Valls ont systématiquement été interpellés, sans effet concret. En tant que président de l'Association nationale des élus du littoral, et parce que je suis très attaché aux territoires ultramarins, j'ai déjà alerté personnellement et directement le ministre Nicolas Hulot sur cette question, par le biais du volet environnemental. Aujourd'hui, malgré les appels au secours des élus mahorais et de la population, le Gouvernement semble mettre ses pas dans ceux de ses prédécesseurs. Ce département français a des besoins vitaux comme l'accès à l'eau, à l'école, à l'électricité, à l'assainissement, au logement et, surtout, à la sécurité. Les réponses apportées par votre gouvernement, à savoir quelques policiers et gendarmes supplémentaires, un déploiement de la police de proximité et un état-major de lutte contre l'immigration clandestine, On nous annonce même une nouvelle conférence sur l'avenir de Mayotte, alors que les assises des outre-mer souhaitées par Emmanuel Macron sont en voie de s'achever. Pour les Mahorais, vos réponses sont malheureusement techniques, technocratiques et, surtout, dilatoires, alors qu'ils attendent un soutien du Gouvernement, c'est-à-dire un engagement politique fort. L'idée de créer une maternité extraterritoriale traduit la reconnaissance que l'immigration clandestine, insupportable à Mayotte, est à l'origine de cette crise, qui risque de dégénérer. Les habitants ne veulent pas de « sous-mesures » - ce sont leurs propres termes. Ils veulent des actes et des solutions juridiques pour stopper l'immigration clandestine, l'explosion des naissances et le regroupement familial. Mayotte a toujours manifesté son attachement à la France, et elle attend autre chose qu'un discours de plus. Allez-vous, monsieur le ministre,

est due à la différence de niveau de vie entre le département de Mayotte et les Comores toutes proches. Entre l'île d'Anjouan et Mayotte, il y a Or la différence de niveau de vie est de 1 à 13. Nous assistons donc à une immigration massive, assortie de difficultés pour les Mahorais, en particulier d'une insécurité grandissante. Et nous avons connu, ces derniers jours, une révolte de la population, incarnée par les élus, mais aussi par l'intersyndicale. Donc oui, nous allons apporter des réponses concrètes à des problèmes qui sont extrêmement graves ! Quand ? J'ai commandé, en début d'année, de nouveaux bateaux, de manière à pouvoir lutter contre l'immigration à Mayotte. Ils seront livrés pendant l'été. En attendant, nous avons demandé qu'un patrouilleur de la marine nationale puisse venir sur les lieux. Le dialogue est engagé avec les élus, parce que c'est avec eux que nous voulons construire un nouvel avenir pour Mayotte dans la République française

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Jeudi dernier, le président des États-Unis a annoncé, de manière unilatérale, la mise en oeuvre de nouvelles barrières douanières. En imposant des taxes de 25 % sur les importations d'acier et de 10 % sur celles d'aluminium, Donald Trump lance une véritable guerre commerciale à l'encontre du reste du monde. Les réactions en Europe ou en Chine ont été immédiates et virulentes. En effet, nous ne pouvons accepter qu'un partenaire commercial lance un conflit international et de nouvelles mesures sans aucune concertation. L'Union européenne a d'ores et déjà annoncé une forme de réplique, en exprimant sa volonté de taxer en retour des produits américains comme le beurre de cacahuète ou les motos Harley-Davidson. Ces symboles peuvent certes marquer les esprits, mais ils ne sont pas à la hauteur des niveaux d'échanges commerciaux qui prévalent dans le cas de l'acier ou de l'aluminium. Pensez-vous, monsieur le ministre, que l'Europe doive entrer dans une surenchère des produits taxés ? Imaginez-vous vraiment que les dernières annonces soient réellement à la hauteur de l'enjeu ? Trois jours après la décision de M. Trump, les États-Unis annonçaient des exceptions possibles pour les produits venant du Canada ou du Mexique, sous condition de nouvel accord commercial.

Nous ne serons forts qu'en étant unis au niveau européen. Il y va de notre développement économique et de l'apaisement des relations commerciales internationales.

La France regrette profondément ces mesures, qui sont des mesures unilatérales. Elles auront un impact négatif sur nos entreprises, que ce soit directement, par le relèvement des droits de douane, ou indirectement, par le choc à la baisse du prix mondial de l'acier et de l'aluminium. Mais, au surplus, la raison invoquée par les autorités américaines invoquée par les autorités américaines pour justifier cette posture, à savoir l'argument de la sécurité nationale, ne nous paraît ni crédible ni étayée. Ces mesures sont d'autant plus regrettables qu'elles pourraient frapper les pays qui, eux, respectent les règles du commerce international et ne sont pas responsables des surcapacités dans le secteur de l'acier et de l'aluminium. Le Président de la République s'est entretenu sur ce sujet, ce week-end, avec le président Trump. Il lui a fait part des observations critiques que je viens d'évoquer. Il faut aujourd'hui une réponse européenne-

la position et l'action de l'Union européenne doivent être à la fois fortes et unies. Tel sera l'enjeu des prochaines semaines : nous doter de la capacité de riposte nécessaire.

». Nous, Européens, sommes en situation de lui dire qu'il s'agit d'une double erreur. L'expérience historique nous a appris que les guerres commerciales ne sont pas bonnes- tout le monde sera perdant, le consommateur américain et les entreprises américaines. Les guerres commerciales débouchent sur le protectionnisme, le nationalisme et, malheureusement, dans certains cas, la guerre. Pourtant, Donald Trump a raison sur un point : la surproduction mondiale et surtout chinoise d'acier dure depuis trop longtemps, et nous avons eu tort de le tolérer. L'une de mes questions est

devons-nous porter ce différend devant l'OMC ? Telle serait la méthode « normale », mais vous savez que les Américains, en refusant de nommer les juges des autorités de règlement des différends, ont paralysé l'OMC. L'OMC n'existe plus de façon active. Enfin, le président Trump a invoqué la sécurité nationale. On peut évidemment se demander en quoi l'Union européenne menace la sécurité nationale des États-Unis.

propos, pour constater avec vous, d'abord, étape après étape, décision après décision, le retrait américain de l'ensemble des forums multilatéraux internationaux.

le retrait. Un nouvel acte en est ici posé. Il est très pénalisant, puisque l'Union européenne est le deuxième exportateur de produits sidérurgiques vers les États-Unis, après le Canada.

Et si, d'aventure, les mesures annoncées devaient être mises en oeuvre, nous devrions, au niveau européen, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires à la défense de nos intérêts industriels.

des participations de l'État dans plusieurs grandes entreprises relevant de secteurs d'activité forts différents, mais toutes d'intérêt national. Je souhaite interroger le Premier ministre au sujet de l'avenir de l'une d'entre elles en particulier, très importante pour le Val-d'Oise. Il s'agit d'Aéroports de Paris, ADP, et de son vaisseau amiral Roissy-Charles de Gaulle. Au vu des enjeux financiers, forts de l'expérience de la privatisation des sociétés d'autoroutes, comment peut-il justifier le calcul court-termiste qui, pour un gain immédiat, prive pour toujours l'État des dividendes importants et dynamiques versés par ADP- 130 millions d'euros en moyenne sur les trois dernières années, soit plus de la moitié des recettes qui seraient issues du « fonds Le Maire » pour l'innovation ? Au vu des impératifs de sécurité nationale, comment peut-il justifier la perte par l'État de la maîtrise directe de la frontière aéroportuaire de Roissy ? Au vu des enjeux régionaux de transports et d'emploi, et après le précédent fâcheux, voulu par Emmanuel Macron, de la cession de l'aéroport de Toulouse, comment l'État compte-t-il associer les collectivités locales concernées ? Au vu des enjeux pour les populations riveraines exposées au bruit, comment M. le Premier ministre peut-il garantir le respect de l'intérêt général dans le cadre de la privatisation de l'activité ? Enfin, après la gestion désastreuse du projet de Notre-Dame-des-Landes, peut-il nous assurer que, dans le dossier ADP, l'État ne sera pas l'otage du résultat de ses propres turpitudes envers le groupe Vinci ? Le Sénat s'était d'ailleurs opposé à sa volonté d'endetter l'État, à rebours de toute logique, pour lancer la réalisation du Charles-de-Gaulle Express, dossier dans lequel le groupe Vinci pourrait obtenir de puissants avantages, alors même qu'il se déclare candidat au rachat d'ADP. Bravo ! La parole

Monsieur le sénateur Arnaud Bazin, le Gouvernement- la presse s'en est fait l'écho -souhaite faire évoluer son portefeuille de participations, afin d'arrêter d'immobiliser l'argent des Français au capital d'entreprises où il n'est pas absolument nécessaire, donc là où le secteur privé est en mesure d'apporter ses financements là où la présence de l'État au capital n'est pas indispensable pour garantir que les intérêts de la France et des Français soient bien respectés, parce qu'il existerait d'autres leviers de régulation qui peuvent permettre de s'en assurer. Il s'agit de trouver des marges pour les investir dans des investissements d'innovation, afin de préparer la croissance de demain. Le groupe Aéroports de Paris, que vous avez cité, monsieur le sénateur, est inclus dans les réflexions, lesquelles sont en cours, mais ne sont pas achevées. Les décisions que vous présentez comme prises ne le sont pas. Je tiens toutefois à vous assurer que, quoi qu'il en soit, nous sommes très attentifs à la défense de l'intérêt des Français sur le long terme. Le cas échéant, et uniquement le cas échéant, le Gouvernement veillerait, bien entendu, à ce que soient mises en place les dispositions nécessaires pour garantir que, s'il n'était plus présent au même niveau au capital d'ADP, une régulation adaptée des aéroports parisiens serait instaurée, afin de s'assurer que la principale porte d'entrée du territoire français continue de fournir un service de qualité, respectueux de toutes les parties prenantes, avec des garanties adaptées en termes notamment de sécurité publique. Vous avez conclu, monsieur le sénateur, en souhaitant que le Gouvernement puisse associer les collectivités locales, les acteurs territoriaux, à la réflexion. Je suis convaincu que, le cas échéant, si cette décision devait être prise, le ministre de l'économie et des finances veillerait à donner suite à votre demande. Nous verrons Merci, monsieur le secrétaire d'État. Vous avez certainement lu le communiqué de presse des sept départements d'Île-de-France unis et de la région d'Île-de-France qui demandent à être entendus, en effet, sur cet aspect stratégique des décisions que vous avez à prendre. Nul doute que nous serons amenés à discuter de nombreuses fois, à de nombreuses étapes de l'avancée de ce

Deux plans Maladies rares se sont succédé depuis 2005, permettant des avancées significatives dans la connaissance de ces pathologies et dans la prise en charge des patients. Ces avancées reposent principalement sur 363 centres de référence, répartis en 23 filières, bénéficiant de financements dédiés. Madame la ministre, votre ministère, au cours du deuxième semestre 2017, a alloué 45 millions d'euros aux nouveaux centres labellisés. Ces crédits fléchés transitent par les budgets généraux des établissements hospitaliers qui hébergent ces 363 centres de référence. 23 professeurs de médecine responsables de ces centres de référence, ainsi que des associations de patients atteints de maladies rares,

de ces crédits. Un tel dysfonctionnement est profondément dommageable pour les patients atteints de maladies rares. Madame la ministre, que répondez-vous aux médecins et aux associations de patients atteints de maladies rares, à la veille du lancement du troisième plan Maladies rares ? ? Quelles mesures envisagez-vous de prendre pour remédier à l'opacité qui entoure l'utilisation effective de ces crédits, pourtant alloués, à l'origine, à une si noble cause ?

merci de votre question, qui permet de mettre en lumière cette difficulté que ressentent nos 3 millions de compatriotes atteints des 6 000 à 7 000 maladies rares recensées.

à la labellisation de 23 filières de santé « maladies rares », qui s'appuient sur 387 centres de référence, 1 800 centres de compétences, avec un budget fléché.

Nous en avons fait l'annonce lors de la Journée internationale des maladies rares, le 28 février dernier. Je tiens d'ailleurs à rappeler qu'une large concertation est menée sur ce sujet, avec six axes prioritaires : assurer au patient un diagnostic plus rapide ; structurer les bases de données pour améliorer la recherche renforcer le rôle des filières pour coordonner les actions des multiples acteurs ; rendre les parcours plus lisibles pour les patients et leurs familles ; renforcer l'innovation, l'objectif européen étant que l'on dispose de 200 nouveaux médicaments d'ici à 2020 ; mettre en place de nouveaux dépistages néonataux. Vous le voyez : nous sommes pleinement mobilisés et nous travaillons sur ces questions budgétaires, afin que les ressources allouées parviennent, évidemment, dans les centres labellisés. La parole

élus et organisations représentatives des salariés se mobilisent pour s'opposer à la remise en cause du modèle hydro-électrique français. Cette ouverture à la concurrence serait d'autant plus stupéfiante que les opérateurs étrangers, européens ou non, pourraient récupérer la gestion d'ouvrages hydro-électriques en France alors que l'inverse n'est pas possible dans la plupart des pays européens. Dois-je rappeler que les barrages constituent des biens nationaux, dont la construction et l'entretien ont été financés par nos concitoyens ? Dois-je rappeler qu'il s'agit d'un produit de première nécessité, l'électricité ? Au-delà des questions de concurrence, faut-il aussi rappeler que nous touchons là à des enjeux de service public de gestion des multiples usages de l'eau ? L'impact du changement climatique devrait nous le rappeler !

Dans un tel contexte, je rappelle que le Gouvernement peut utiliser la procédure de prolongation des concessions contre investissements, que nous avons fait adopter dans la loi relative à la transition énergétique des informations circulent selon lesquelles le Gouvernement se serait engagé sur un premier calendrier de mise en concurrence de lots en regroupements barycentriques, mais aussi sur un dispositif qui conduirait à empêcher- je n'ose le croire ! -les opérateurs historiques de remporter toutes les concessions, quand bien même leurs offres seraient les meilleures. Monsieur le ministre, que valent donc ces informations ? Le Gouvernement a-t-il l'intention de se battre sur ce dossier, notamment en utilisant la procédure de prolongation des concessions contre travaux et investissements ?

ai-je besoin de rappeler- vous l'avez fait -que l'hydroélectricité est un pilier de la transition énergétique ? Cette énergie est au coeur de nos territoires et, entre autres, participe à la bonne gestion des ressources en eau. Vous l'avez dit : voilà maintenant dix ans que la Commission européenne a demandé l'ouverture à la concurrence des concessions hydro-électriques. Le droit français, qui est conforme au droit européen, prévoit à ce titre que les concessions hydro-électriques échues doivent être renouvelées par une mise en concurrence.

et d'assurer, autant que faire se peut, un partage équilibré des bénéfices au profit des territoires. En outre, les concessions peuvent être regroupées pour faciliter leur exploitation et favoriser la sûreté. Enfin, il existe un mécanisme- vous l'avez évoqué, monsieur le sénateur -qui ouvre la possibilité d'une prolongation contre travaux, dans le respect de la directive Concession. Par ailleurs, s'agissant des questions dont vous vous faites l'écho, et que les journaux ont relayées encore ce matin, en lien avec le mouvement social, je tiens à vous rassurer : le statut des personnels sera dans tous les cas de figure préservé, et les cahiers des charges devront évidemment prévoir la reprise des personnels par le nouvel exploitant. Ce n'est pas la question ! Il ne s'agit pas, contrairement à ce que j'ai lu, d'une privatisation. Je vous confirme en effet que les barrages vont rester la propriété de l'État, notamment pour en garantir la sécurité. En aucun cas la mise en concurrence ne devra se traduire par un déficit de sécurité. Vous nous demandez si nous sommes montés au front, et si nous continuons à défendre la position française. Je l'ai fait à plusieurs reprises à Bruxelles ; nous avons également reçu la commissaire au ministère. La France va continuer à défendre

La séance est reprise. Les conclusions de la conférence des présidents réunie ce jour et complétant l'ordre du jour établi par la réunion de la conférence des présidents du 21 février 2018 sont consultables sur le site du Sénat. Je vous informe notamment que la conférence des présidents a décidé de déplacer les questions au Gouvernement initialement prévues le jeudi 22 mars au mardi 20 mars, à seize heures quarante-cinq, à l'issue du scrutin solennel sur le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observations d'ici à la fin de la séance. à 16 heures - Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour un État au service d'une société de confiance

loi. Notre position sur cette annexe reste celle que nous avons exprimée dans notre rapport et lors de l'examen du texte en commission. Si personne ne peut contester le bien-fondé des principes et objectifs qui y sont présentés, force est de constater qu'ils sont bien trop nombreux pour être de véritables principes généraux, clairs et lisibles. Nous constatons également que cette annexe est dépourvue de portée normative ; nous nous interrogeons toujours, à ce titre, sur son utilité réelle. Nous défendons donc une position de compromis : globalement favorables aux principes qui figurent dans cette annexe, nous ne souhaitons pas la supprimer, mais, ayant de très profonds doutes sur son utilité réelle, nous ne pensons pas nécessaire de la modifier.

de courtoisie des usagers semble en dehors du champ de la stratégie nationale, qui ne liste que des objectifs à destination de l'administration et de ses agents.

De la même manière, s'agissant de l'amendement n° 111 de notre collègue François Patriat, le principe d'autonomie qu'il défend semble déjà présent au quatrième alinéa de l'annexe visée. de l'amendement n° 165 d'Élisabeth Lamure, tendant à conditionner l'entrée en vigueur d'une norme nouvelle applicable aux entreprises à la suppression d'une norme préexistante, semble poser un problème de constitutionnalité. Il s'agit en effet d'un principe ayant une véritable portée normative, mais qui restreint le champ de la loi et des règlements tels qu'ils sont respectivement définis aux articles 34 et 37 de la Constitution. Comme je l'ai dit, la commission demande

les grandes orientations définies dans la stratégie nationale d'orientation de l'action publique. Toutefois, la rédaction que vous nous proposez paraît oublier certaines orientations qui, à nos yeux, sont essentielles, s'agissant notamment de l'évaluation de l'action publique, de la conception de son efficacité en termes de délais et de coûts, ou encore de la dématérialisation.

nous reprenons à notre compte les arguments de Mme la rapporteur. Le respect et la courtoisie semblent devoir s'imposer à tous- ce serait l'idéal ; ce n'est, effectivement, pas toujours le cas. De notre point de vue, si l'administration doit faire preuve de savoir-vivre à l'égard des usagers,

proposition de loi constitutionnelle prévoyant déjà d'assortir toute mesure législative de charges nouvelles de la suppression de charges équivalentes. Nous étions bien dans le même

Il s'agit donc de traiter le volet simplification et réduction des délais administratifs dans le cadre exhaustif et cohérent des textes sectoriels. Quel est l'avis de la commission l'avis de la commission spéciale ? Cet amendement tend à préciser que les dispositions visant à réduire les délais administratifs ne doivent être prises que dans des textes sectoriels et que chaque texte sectoriel doit en comporter. Je partage la volonté de ne prendre que des mesures adaptées à chaque secteur concerné pour éviter l'éclatement des problématiques. Mais nous constatons que l'amendement présenté pose des problèmes, notamment d'ordre constitutionnel j'en suis désolée, madame Lamure. Pour les dispositions réglementaires applicables en matière de droit des entreprises, l'adoption de cet amendement aurait pour conséquence de restreindre le champ du pouvoir réglementaire tel qu'il est défini à l'article 37 de la Constitution, ce qui semble inconstitutionnel. Pour ce qui est des dispositions législatives, l'amendement serait inopérant, puisque n'importe quelle loi postérieure pourrait y déroger. La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l'avis serait défavorable. Quel est

d'un vrai changement dans la conception entre les citoyens et l'administration. C'est l'idée que l'on peut évidemment commettre une erreur de bonne foi.

La législation encadrant leur situation et leur statut est particulièrement complexe. Elle fait intervenir le droit français, le droit suisse, ainsi que le droit international et européen. sont donc, par nature, exposés à un risque élevé de commettre des erreurs dans leurs rapports avec les administrations françaises. La ministre des solidarités et de la santé a d'ailleurs porté devant la Cour de cassation une procédure pour statuer sur les conflits d'affiliation aux organismes de sécurité sociale ; nous attendons sous peu l'arrêt de la Cour. nouveau droit à l'erreur, permettez-moi d'espérer que les frontaliers bénéficieront de toute la bienveillance de l'administration et que la recherche de solutions amiables guidera plus que jamais à l'avenir l'action des services concernés par ces questions techniquement complexes, mais qui plongent les personnes dont il s'agit dans des situations humainement inacceptables. La parole

Notre prix Nobel d'économie Maurice Allais fustigeait déjà en 1977 le « pouvoir réellement exorbitant des administrations technocratiques », en regrettant que la fiscalité « échappât au contrôle démocratique du Parlement Nous sommes désormais face à l'extrême complexité du maquis fiscal, source d'insécurité juridique. Qui veut s'en convaincre n'a qu'à consulter ces énormes volumes ! Et encore : je n'en ai amené qu'un échantillon ; il faudrait faire de la musculation pour pouvoir tous pouvoir tous les porter ! Afin de ne pas faire d'erreur, un contribuable peut solliciter l'administration fiscale pour valider un montage. L'administration a trois mois pour répondre. Si elle ne le fait pas, cela n'a aucune conséquence. Le problème reste entier pour le contribuable. J'avais proposé un amendement pour le résoudre : si l'administration fiscale ne répondait pas au bout de trois mois, comme prévu par les textes, cela valait accord ; le contribuable pouvait alors agir en confiance et en sécurité. Mon amendement a été déclaré irrecevable au motif que son adoption « créerait une contrainte supplémentaire pour l'administration qui n'est pas absorbable à effectif constant ». Il ne sera donc pas discuté en vertu de l'article 40 de la Constitution, et au prétexte que son adoption créerait une charge supplémentaire pour l'État. énième atteinte à l'exercice du droit d'initiative parlementaire et au principe de la légalité fiscale, qui, par application de l'article XIV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, voudrait que le Parlement dispose d'une compétence exclusive en matière fiscale. fiscale. Si je vous suis bien, vous n'avez pas assez d'effectifs pour répondre dans les trois mois aux contribuables qui vous sollicitent, mais vous en avez suffisamment pour les contrôles fiscaux ! Vous en avez même tellement que vous proposez de vous limiter à neuf mois de contrôle fiscal pour une PME tous les trois ans. et un ans d'exercice au Royaume-Uni, je n'ai eu qu'un contrôle pour ma PME, et il a duré une journée ! Pour créer une société de confiance, il aurait fallu que l'État choisisse de prévenir les erreurs plutôt que de les provoquer en entretenant une fiscalité incompréhensible. Ce que nous faisons actuellement ici ne saurait créer les conditions d'une société de confiance. Cela participe plutôt au harcèlement textuel qui alimente une société de défiance.

usages. Le projet de loi prévoit une série d'exceptions à la règle. Ainsi en est-il du droit de l'Union européenne ou de la sécurité des personnes et des biens. Par cohérence avec l'état actuel du droit, nous proposons d'ajouter à la liste des infractions n'ouvrant pas droit à l'exercice du droit à l'erreur celles qui concerneraient les atteintes, parfois commises de manière intentionnelle, aux droits tout à fait élémentaires des salariés. Il est vrai que les avancées en matière de droit du travail ont été pour le moins limitées ces derniers temps Prenons un exemple concret : un exploitant agricole n'aurait ainsi pas le droit à l'erreur quand il s'agirait de remplir un dossier de subvention au titre de la politique agricole commune, mais il pourrait être considéré comme fautif de bonne foi pour peu qu'il ait omis de déclarer correctement quelques-uns des travailleurs saisonniers qui l'auraient aidé, par exemple pour la récolte. Quel est

En réalité, il est satisfait par le droit existant eu égard à la hiérarchie des normes, comme cela a été indiqué lors des débats en commission. Le droit international prime en effet le droit national sans qu'il soit nécessaire de l'expliciter, et il en va de même pour les dispositions législatives d'ordre public, auxquelles il ne peut pas être dérogé. En conséquence, les dispositions relatives au droit à l'erreur ne s'appliquent pas lorsque des obligations résultant d'une convention internationale s'y opposent, par exemple en matière de droit du travail. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons supprimé à ce même article 2, pour le droit au contrôle, une référence inutile au respect des conventions internationales.

Le présent projet de loi exclut de l'application du droit à l'erreur les règles issues du droit européen. Or, dans le cas de la politique agricole commune, la PAC, il existe plusieurs volets qui sont définis par les États membres. Chaque année, pour bénéficier des aides financières européennes de la PAC, les agriculteurs doivent remplir des dossiers de demande rédigés par notre administration et nos services français dans lesquels il n'est pas rare de se perdre. Les nouveaux dispositifs de la PAC impliquent des dossiers de plus en plus complexes, et les formulaires demandent un haut degré de précisions. Le travail quotidien de nos agriculteurs est rude, prenant. Vous le savez, ils n'ont aujourd'hui ni forcément le temps ni l'appui technique pour remplir ces dossiers. Cet amendement vise donc à considérer que, pour ces volets définis par les États membres, en l'occurrence ceux qui relèvent des décisions de l'État français, le droit à l'erreur peut s'appliquer. Pouvez-vous nous confirmer que, s'il est prouvé qu'il s'agit d'une procédure française, établie par le pouvoir réglementaire ou législatif, le droit à l'erreur s'applique pour l'agriculture comme pour toute autre activité ? Quel est l'avis de la commission spéciale ? Cet

ce qui recouvre les hypothèses dans lesquelles l'administration est tenue de prononcer une sanction sans disposer d'une marge d'appréciation, faute de quoi elle méconnaîtrait une obligation qui lui incombe en vertu du droit de l'Union européenne. À cet égard, concernant la politique agricole commune, et comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi, le droit européen procède à une harmonisation des contrôles et des sanctions, les États membres ne disposent ainsi d'aucune marge d'appréciation dans l'application des sanctions.

pour l'application desquelles la France ne dispose pas de marge d'appréciation pour prononcer la sanction. Par conséquent, pour les agriculteurs, que vous évoquez, c'est seulement lorsque l'État membre n'a pas d'autre choix que d'infliger une sanction au titre de la politique agricole commune que le droit à l'erreur ne s'applique pas. En revanche, chaque fois que les États membres disposent d'une marge d'appréciation dans le prononcé d'une sanction, les agriculteurs pourront faire jouer leur droit à l'erreur. J'ajoute que cette exception vaut pour la PAC, comme pour toute autre réglementation européenne.

les exceptions au droit à l'erreur sont limitées par l'article 2 à la méconnaissance de règles préservant directement la santé publique, l'environnement ou la sécurité des personnes ou des biens. Comme je l'ai indiqué lors de l'examen du texte par la commission spéciale, il me semble que l'exclusion du champ du droit à l'erreur d'atteintes directes à ces règles permet à la fois de préserver ces intérêts fondamentaux tout en encadrant le champ des exceptions. En conséquence, seules les atteintes directes à l'environnement sont exclues du droit à l'erreur. L'adoption du présent amendement reviendrait à prévoir des exceptions aux exceptions au droit à l'erreur en matière d'environnement, ce qui ne me paraît pas pertinent. Par ailleurs, les dispositions du code de l'environnement visées ne pourraient pas forcément entrer dans le champ d'application du droit à l'erreur, qui ne concerne que les procédures dans lesquelles les usagers sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction pécuniaire ou d'une suspension de prestation. Par exemple, le paragraphe I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement prévoit une procédure de mise en demeure de respect des règles du code, dont des dispositions en cas d'urgence visant à prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement, qui seraient de toute façon exclus

partage l'avis de la commission. L'amendement proposé vise à étendre l'application du dispositif transversal sur le droit à l'erreur aux sanctions appliquées dans le cadre du code de l'environnement. Les articles de police dont il est question sont transverses à tout le code de l'environnement et ne s'appliquent pas qu'aux installations classées Or ces articles permettent aux sanctions en matière d'environnement d'être effectives et conformes aux exigences européennes tout en préservant la possibilité de régularisation par l'administré concerné.

sans réellement présenter d'intérêt pour les exploitants de bonne foi, qui peuvent déjà régulariser leur situation sans encourir de sanction après la mise en demeure. La

le Conseil d'État estime, de son côté, qu'en créant une procédure supplémentaire sans simplifier les normes et les procédures existantes, le mécanisme du droit au contrôle ne répond que très imparfaitement à cet objectif. Ce dispositif, dont le champ d'application est extrêmement vaste, pourrait porter atteinte au bon fonctionnement de l'administration, dès lors qu'il prévoit que celle-ci est tenue de faire droit à cette demande dans un délai raisonnable, sans tenir suffisamment compte de ses moyens et effectifs. relève que les moyens des services de l'État ont souvent été fortement réduits et ne leur permettent pas toujours d'assumer leurs missions premières, au risque d'exposer la responsabilité de l'État, ainsi que celle de ses agents

Je souscris comme vous, mon cher collègue, aux arguments du Conseil d'État que vous évoquez et que j'ai d'ailleurs relevés dans le rapport de la commission spéciale, à savoir le manque de précision des dispositions proposées et l'absence de véritable étude de leur impact. Toutefois, nous n'avons pas proposé de supprimer ce dispositif, dans la mesure où nous partageons l'objectif final de simplifier les relations des usagers avec l'administration dans le respect du droit. La commission spéciale a d'ailleurs adopté deux amendements en ce qui concerne le droit au contrôle. En premier lieu, elle a fixé un délai maximum de six mois dans lequel l'administration doit procéder au contrôle, afin de rendre le dispositif plus attractif et opérationnel. Si une entreprise ou un particulier souhaite bénéficier d'un contrôle, c'est afin de sécuriser sa situation juridique dans les meilleurs délais. L'administration pourra d'ailleurs toujours refuser le contrôle de façon discrétionnaire, s'il conduit à compromettre son bon fonctionnement. En second lieu, la commission spéciale a souhaité sécuriser l'opposabilité des conclusions expresses rédigées par l'administration à l'issue du contrôle, en prévoyant qu'elles ne sont opposables que si elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, reprenant une formulation de l'article 4 du projet de loi.

Mon cher collègue, votre souhait est pleinement satisfait par l'article, puisque, comme nous l'ont confirmé tant la direction de la sécurité sociale que les responsables de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ce dispositif, dit de visite-conseil, est légalisé par le droit au contrôle, qui s'appliquera bien dans le champ des contrôles opérés par l'URSSAF.

Le présent amendement inclut à l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration les enquêtes de satisfaction des usagers de l'administration parmi les documents devant être rendus publics par cette dernière. Si j'adhère tout à fait à l'objectif de mesure des résultats de l'administration, notamment grâce à l'évaluation de la satisfaction des usagers- démarche qui nous avait d'ailleurs été présentée par la direction interministérielle de la transformation publique -, cet amendement m'apparaît satisfait par le droit en vigueur. En effet, les administrations concernées doivent déjà publier ces enquêtes de satisfaction, puisqu'elles rentrent dans le champ d'application du 4° de l'article L. 312-1-1, que l'amendement veut modifier. En effet, il s'agit bien de données « dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental

En faire bénéficier les collectivités locales au même titre que les usagers brouillerait l'objectif clairement affiché de cette réforme, qui s'adresse aux usagers dans leurs relations avec toutes les administrations, et non aux relations entre administrations elles-mêmes qui ne peuvent pas être mises sur le même plan. Par ailleurs, on pourrait aussi se demander pourquoi ce droit ne serait étendu qu'aux relations entre l'État, entendu au sens large, et les collectivités territoriales, et pas aux relations entre collectivités territoriales elles-mêmes. De la même manière, rien ne nous paraît justifier que ce droit à l'erreur ne s'exerce qu'au profit des collectivités territoriales, et non pas également à celui de l'État.

En effet, tout comme les usagers, les collectivités territoriales et leurs groupements ont aussi besoin du regard bienveillant de l'État et des organismes de sécurité sociale dans le cadre des missions qu'ils doivent accomplir au quotidien et des procédures qu'ils doivent engager dans des conditions parfois difficiles. Je ne considère pas que cette mesure risquerait de diluer le dispositif initial, dans la mesure où elle s'appliquerait dans les mêmes conditions que celles de l'article 2, c'est-à-dire dans les hypothèses où les collectivités territoriales sont, de fait, dans la situation d'usagers de l'administration de l'État ou des organismes de sécurité sociale. Typiquement, je pense aux demandes de subventions. Par ailleurs, si effectivement le rôle de conseil des préfectures auprès des collectivités territoriales est indispensable, les services de l'État n'ont plus forcément les moyens d'apporter l'appui juridique et l'expertise suffisants, notamment aux plus petites communes, qui sont souvent démunies

cette disposition pourrait s'appliquer, je l'encourage chaudement à venir dans un département rural comme le mien, où il n'y a plus de trésorerie, où les sous-préfectures ne sont pas ouvertes aux élus, où on règle à peu près tout par téléphone

Par cet amendement, je souhaite éviter que le droit à régularisation en cas d'erreur soit privé de son effectivité dans le domaine social. Comme l'a souligné le Défenseur des droits dans son avis sur le présent projet de loi, il existe un risque que le nouvel article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'impose pas aux organismes de prestations familiales ou d'assurance vieillesse. Le code de la sécurité sociale prévoit en effet une règle spécifique s'agissant de l'erreur des assurés, une règle d'ailleurs moins favorable puisqu'elle assimile erreur et fraude. Vous le savez, le code des relations entre le public et les administrations régit les relations entre le public et les administrations, y compris les organismes sociaux, « en l'absence de dispositions spéciales applicables ». Le risque est donc réel que les dispositions spéciales du code de la santé publique l'emportent sur la règle générale du droit à la rectification en cas d'erreur. Pour éviter cette incertitude qui serait gravement préjudiciable à la quasi-totalité de nos concitoyens, je vous propose d'introduire la règle du droit à l'erreur dans l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Quel est l'avis de la commission spéciale ? la commission spéciale ? Cet amendement tend à ce que le droit à l'erreur soit appliqué dans les relations entre les organismes de sécurité sociale et les bénéficiaires de prestations, dans les cas où ces derniers s'exposent à des sanctions en raison de déclarations erronées. J'ai pris l'attache de la Caisse nationale des allocations familiales et de la direction de la sécurité sociale, qui m'ont indiqué que, dans les faits, aucune pénalité n'est aujourd'hui appliquée en cas d'erreur de bonne foi. L'objectif des auteurs de l'amendement semble donc satisfait, mais la commission spéciale a souhaité demander au Gouvernement son avis sur cet amendement. Quel est l'avis du Gouvernement l'avis du Gouvernement ? Cet amendement vise à restreindre le prononcé de pénalités financières aux cas de fraude pour les branches vieillesse et famille. Le Gouvernement partage le souhait des auteurs de l'amendement de limiter les pénalités aux personnes manifestement de mauvaise foi ou qui fraudent. Bien que la situation soit extrêmement rare, comme l'a rappelé Mme la rapporteur, le fait de l'inscrire dans la loi permettra de l'acter de manière définitive et solide. C'est pourquoi l'avis du Gouvernement est favorable sur cet amendement.

de l'évaluation des voies et moyens annexé à la loi de finances laisse apparaître que, même quand une entreprise ou un particulier se trouve engagé dans un processus de redressement fiscal, il n'est pas rare que des allégements soient opérés sur la facture. Ainsi, l'examen précis des situations concrètes des particuliers comme des entreprises peut fort bien amener l'administration à transiger et à atténuer ici les pénalités, ailleurs les sommes dues au titre de l'intérêt de retard. Ces comportements de l'administration procèdent de la doctrine fiscale, établie non seulement par la loi, aussi par l'importante production réglementaire de ces administrations- décrets, circulaires ... -, et veillent, qu'on le croie ou non, à tenir effectivement compte des capacités contributives du redevable. Les recours gracieux, cela existe toujours, sans parler des abandons de pénalité

: La parole est à Mme Gisèle Jourda. En 2017, le paiement par prélèvement automatique ou en ligne est devenu obligatoire pour tout avis d'impôt supérieur à 2 000 euros. Le seuil de paiement obligatoire sera abaissé à 1 000 euros en 2018 et à 300 euros en 2019. Cependant, nul n'ignore sur ces travées

Ainsi, en plus de nuire considérablement à l'attrait et au développement de ces territoires souvent ruraux, il se trouve- vous en conviendrez -que plusieurs des habitants de ces zones ne peuvent bénéficier d'une connexion suffisante pour procéder à la gestion de leurs impôts par internet. Vous me direz que, s'ils en informent l'administration, ils peuvent toujours utiliser la déclaration papier. Je vous réponds que, si on peut protéger en amont nos concitoyens de toute sanction injuste de l'administration qui viendrait pénaliser ceux qui vivent dans ces zones, en reportant l'obligation de télédéclaration et surtout celle de télépaiement à 2025, c'est beaucoup mieux.

Premièrement, l'obligation de déclarer l'impôt sur le revenu en ligne n'est pas applicable aux contribuables qui ne disposent pas d'un accès à internet. Deuxièmement, les contribuables qui estiment ne pas être en mesure de faire leur déclaration en ligne, pour une raison ou une autre et pourvu qu'ils en informent l'administration, peuvent toujours utiliser la déclaration papier. Il est toujours possible d'aller plus loin, mais se pose alors la question du critère à retenir. Or il n'existe pas de définition de la « zone blanche » : s'agit-il de la 4G ou du très haut débit ? Comment définir strictement ces zones, sachant qu'elles évoluent en permanence et qu'elles sont différentes en fonction des opérateurs ? Pour mémoire, la déclaration en ligne de l'impôt sur le revenu est maintenant obligatoire pour tous les contribuables dont le revenu dépasse 15 000 euros deviendra obligatoire en 2019 pour l'ensemble des contribuables disposant d'un accès à internet. À défaut, une amende de 15 euros par déclaration est appliquée. En conclusion, la commission émet un avis de sagesse

que la résidence principale des contribuables est équipée d'un accès à internet. Dans ce cadre, le dispositif législatif comporte déjà une exemption de l'obligation de déclarer en ligne pour les usagers dont la situation, l'âge, le handicap, l'accès au numérique, soit par non-équipement, soit par mauvaise maîtrise du numérique ou par couverture insuffisante, ne leur permettent pas de déclarer en ligne. Ainsi, l'article 1649 B du code général des impôts prévoit que ceux qui estiment ne pas être en capacité de déclarer en ligne peuvent utiliser une déclaration papier, sans autre démarche spécifique. La direction générale des finances publiques informe et rassure les usagers quant à cette exemption au moyen d'une mention visible sur la première page de la déclaration des revenus. S'agissant de l'amende forfaitaire de 15 euros

En outre, l'adhésion au prélèvement à l'échéance mensuelle peut être faite par courrier, mail ou téléphone auprès des centres prélèvement service. Ces modes de souscription répondent complètement aux difficultés que pourraient rencontrer certains usagers, notamment la fracture numérique, le grand âge ou des situations de handicap. Enfin, les services territoriaux de la DGFiP ont pour consigne d'accompagner les usagers en difficulté qui se présenteraient aux guichets pour faciliter leurs démarches de paiement dématérialisé. Compte tenu de toutes les dispositions prises pour favoriser l'inclusion de tous les publics, votre amendement nous paraît donc satisfait. Les exceptions déjà prévues par le droit vont au-delà des seuls besoins des habitants des zones blanches que vous mentionnez dans votre amendement et prennent en considération d'autres obstacles à la télédéclaration que la seule non-couverture. Espérant vous avoir convaincue et, surtout, vous avoir rassurée,

très haut débit en 2022. Par ailleurs, comme le Président de la République l'a annoncé en décembre dernier lors de la conférence nationale des territoires, 100 % des Français devraient pouvoir disposer, en 2020, d'un débit suffisant

je partage complètement le propos de notre collègue : une société de confiance ne se décline pas uniquement sous l'aspect numérique.

je crois voir naître un rapport de forces, je ne serai pas long, mais je veux simplement attirer votre attention sur le fait que l'exemption de l'obligation de télédéclaration en cas de